La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 7 juin a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025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 Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer en votre nom la présence en tribune officielle d'une délégation du Parlement australien conduite par M. Scott Ryan. La délégation est accompagnée par notre collègue Marc Daunis, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Australie. Cette délégation effectue actuellement un séjour d'étude en France, destiné à renforcer les liens entre nos deux pays. La fraternité d'armes forgée durant la Première Guerre mondiale s'est transformée depuis en une véritable alliance stratégique, comme en témoigne le contrat historique signé entre nos deux pays pour la construction de douze sous-marins australiens par un grand groupe industriel français. Après le déplacement en Australie du Président de la République en mai dernier, ce partenariat se poursuit aujourd'hui dans le domaine de la diplomatie et de la coopération parlementaires. Ainsi, la délégation a été reçue hier par notre collègue Philippe Dallier, vice-président du Sénat en charge des relations internationales et des groupes interparlementaires d'amitié, au nom du président du Sénat, M. Gérard Larcher, qui était en déplacement en province. Elle s'est entretenue ensuite avec M. Robert del Picchia, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le thème de la diplomatie parlementaire. Enfin, la délégation a longuement échangé sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et de cybersécurité. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France lui soit profitable et contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux pays. L'ordre

du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination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

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi soumise à votre examen cet après-midi est singulière à plusieurs égards. égards. Déposée au Sénat le 30 mars dernier par le président Gérard Larcher lui-même et huit présidents de commission, ainsi que par la présidente de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, du contrôle et des études, elle l'a été le même jour à l'Assemblée nationale par le président de celle-ci et quatre présidents de groupe politique. Cette proposition de loi vise à mettre en oeuvre une disposition introduite dans la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique par un amendement de M. le président de la commission des lois, Philippe Bas. Cette disposition prévoit que la participation des sénateurs et des députés aux organismes extraparlementaires, les OEP, et aux instances consultatives est limitée, à compter du 1 juillet 2018, au nom du principe de séparation des pouvoirs, aux cas où leur présence a été prévue par la loi. Le texte dont nous débattons cet après-midi répond à cette nouvelle exigence. Il s'agit, en premier lieu, de simplifier les règles qui régissent la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires. La présence des parlementaires est aujourd'hui prévue au sein de 193 organismes. Pour 112 d'entre eux, cette présence est prévue par la loi ; pour les 81 restants, elle résulte d'un acte réglementaire. Durant les dernières décennies, ces chiffres n'ont cessé de croître. Depuis octobre 2014, pas moins de 58 nouvelles instances ont été créées, dont 29 au cours de la seule année parlementaire 2016-2017. Organismes de décision, de consultation obligatoire, de recueil d'avis ou encore d'évaluation des politiques publiques, les OEP sont multiples. De même, les règles relatives à la nomination des parlementaires varient selon les organismes, ainsi que les objectifs de respect de la parité et du pluralisme en leur sein. L'absence de règles harmonisées est une source de complexité, d'autant que le Sénat et l'Assemblée nationale sont appelés, lors de chaque mandature, à procéder respectivement à plus de 660 et près de 700 nominations. Ces désignations font l'objet de toute l'attention du Gouvernement, qui attache une importance de premier ordre à ce que les organismes extraparlementaires puissent se réunir dans une formation complète pour pouvoir assumer pleinement leur rôle.

Le travail de simplification entrepris par l'Assemblée nationale et que le Sénat, sous l'impulsion de son rapporteur, a souhaité approfondir est essentiel également en ce qu'il vise à permettre aux parlementaires de jouer pleinement leur rôle, là où leur présence et leur expertise sont utiles. L'entreprise de simplification encouragée par cette proposition de loi a été l'occasion d'un inventaire, que je crois exhaustif, de ces organismes extraparlementaires, comme en témoigne le rapport très complet Le Gouvernement et les OEP saisis par le rapporteur se sont prêtés de bonne grâce à un examen de leur activité et de leur contribution aux différentes politiques publiques relevant de leur compétence. C'est toujours un exercice salutaire Ce travail mené par le Gouvernement participe à l'objectif d'une action publique recentrée, plus efficace et plus lisible par nos concitoyens. Cette revue générale, que le rapporteur nous a invités a permis d'identifier tous les OEP au sein desquels la présence des parlementaires lui est apparue nécessaire, comme le Conseil national du bruit. À l'inverse, il s'est montré plus entreprenant que l'Assemblée nationale en matière de simplification du paysage des OEP, puisqu'il a supprimé la présence des parlementaires dans un nombre significatif d'organismes. À cet égard, le Gouvernement regrette le sort réservé au comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative, dont le rapporteur a choisi de confier les compétences au Haut Conseil à la vie associative. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce sujet.

Je précise toutefois que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait rejeté la suppression de l'entrée en vigueur différée de l'ensemble du texte : l'Assemblée nationale a en effet procédé à un renouvellement général des nominations il y a moins d'un an. Je ne doute pas que cette disposition, comme d'autres adoptées par la Haute Assemblée, nourrira un dialogue bicaméral constructif et fécond dans la perspective de la commission mixte paritaire. Je forme le voeu que ce dialogue prospère et que la proposition de loi, à laquelle le Gouvernement est évidemment favorable et qui doit permettre une meilleure participation des parlementaires aux OEP, ainsi qu'une meilleure lisibilité de leur action pour nos concitoyens, puisse être prochainement adoptée de façon définitive. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, comment garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et simplifier les modalités de leur nomination ?

ce texte a été examiné par notre commission des lois selon la procédure de législation en commission. La participation de députés et de sénateurs à des organismes extraparlementaires s'inscrit dans une longue tradition, qui remonte au XIX siècle avec la création de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Les organismes extraparlementaires ont trois objectifs principaux ils renforcent le contrôle de l'action du Gouvernement, améliorent l'évaluation des politiques publiques et permettent aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens. La participation des parlementaires à ces organismes extérieurs est soumise au contrôle déontologique des instances compétentes de chaque assemblée. Rendue publique, cette participation ne donne lieu à aucune rémunération.

Par ailleurs, les organismes extraparlementaires sont désormais tellement divers qu'il est presque impossible d'en établir une typologie cohérente. La situation actuelle pose au moins trois difficultés elle accroît les contraintes, déjà lourdes, qui pèsent sur les agendas des députés et des sénateurs ; elle laisse une grande marge de manoeuvre au pouvoir réglementaire ; elle fait coexister des règles de nomination disparates.

En octobre 2016, le président du Sénat a refusé de désigner des sénateurs pour siéger dans des organismes extraparlementaires de nature réglementaire. Puis, en septembre 2017, le Sénat a adopté, sur l'initiative du président de la commission des lois, un amendement au projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique. Désormais, un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs est énoncé à l'article L.O. 145 du code électoral : à compter du 1 juillet 2018, seule une loi peut ou pourra prévoir la présence d'un parlementaire, député ou sénateur, dans un organisme extraparlementaire. Grâce à ce texte, les procédures de nomination des députés et des sénateurs dans les organismes extraparlementaires ils seront désormais nommés par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, sauf disposition législative contraire. Des règles uniformes seront fixées pour que ces nominations respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes. De même, le principe du pluralisme politique sera consacré dans la loi.

les autres. Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi, qui amplifie les efforts de rationalisation en ce qui concerne la présence des parlementaires dans ces organismes. préparatoires, j'ai tenu à poursuivre les efforts de concertation engagés depuis plusieurs mois par les présidents des deux assemblées, en consultant les présidents de groupe et de commission du Sénat, mais également les organismes concernés. Mes chers collègues,

Je vous propose d'approuver la simplification des modalités de désignation des parlementaires. La proposition de loi doit être adoptée avant le 1 juillet 2018 pour garantir la présence de députés et de sénateurs dans les organismes extraparlementaires que nous pouvons considérer comme étant les plus utiles. En outre, la simplification des règles de nomination dans les organismes extraparlementaires et les garanties apportées en termes de parité et de pluralisme me semblent particulièrement opportunes.

future loi comportera donc des efforts de rationalisation importants, qui iront au-delà de ceux proposés par l'Assemblée nationale. J'ai pu constater l'attachement des parties prenantes

faut aussi éviter le plus possible de pérenniser dans la loi des commissions administratives consultatives qui avaient vocation à être supprimées par le Gouvernement. Seule la présence des parlementaires dans les commissions consultatives les plus essentielles doit être maintenue pour éviter pour éviter un nouvel empilement de structures administratives. Avec les amendements adoptés, nous avons supprimé la présence de parlementaires dans treize structures. Dans la plupart des cas, il s'est agi non pas de supprimer des organismes mis en place

Mes chers collègues, la préoccupation de voir garantie notre présence dans les organismes extraparlementaires a été mise en lumière avec l'examen de ce texte. Au moment où de nouveaux organismes de ce type sont,

Depuis 2016, le président du Sénat refusait, compte tenu de ce qui était considéré comme une atteinte à la séparation des pouvoirs, de désigner des sénateurs dans certains organismes extraparlementaires.

la présence de députés et de sénateurs au sein d'organismes extraparlementaires est une tradition républicaine qui remonte au XIX siècle avec la création de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Les organismes extérieurs au Parlement ont trois missions principales : renforcer le contrôle de l'action du Gouvernement, améliorer l'évaluation des politiques publiques et permettre aux organismes concernés de mieux appréhender les aspirations de nos concitoyens. Le nombre d'organismes extérieurs au Parlement a connu une croissance exponentielle depuis les débuts de la VRépublique, passant de dix-sept en 1958 à deux Les organismes extraparlementaires sont désormais tellement divers qu'il est quasi impossible d'en établir une typologie cohérente. Depuis 2015, le Sénat mène une réflexion sur ces organismes extraparlementaires. Cette réflexion répond à un double objectif : recentrer l'activité des parlementaires sur les travaux de leur assemblée et mettre fin à des pratiques attentatoires au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En effet, aujourd'hui, dans 40 % des organismes concernés, la présence de parlementaires a été prévue par un texte réglementaire, et non par la loi. Cette réflexion engagée par le Sénat a abouti à l'adoption de l'article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui fixe un principe à la fois clair et respectueux de la séparation des pouvoirs à compter du 1 juillet 2018, seule une loi pourra prévoir la présence d'un député ou d'un sénateur dans un organisme extraparlementaire. C'est dans ce contexte qu'une proposition de loi conjointe des présidents des deux chambres du Parlement a été déposée, visant trois objectifs rationaliser les procédures de nomination des députés et des sénateurs au sein des organismes extraparlementaires, garantir leur présence dans les structures où elle paraît justifiée et la supprimer lorsque cette justification a cessé. La commission des lois a prolongé la logique de rationalisation de cette proposition. Ainsi, elle a simplifié l'application du principe de parité pour les nominations dans les organismes extraparlementaires et poursuivi l'harmonisation des modes de nomination. également prévu la désignation de suppléants dans les organismes où cela s'avérerait nécessaire, comme le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale, la commission des lois a supprimé la présence de parlementaires dans treize organismes supplémentaires. À l'inverse, elle l'a prévue pour le Conseil national de l'air et le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Au total, la présence de parlementaires serait maintenue au sein de cent soixante-quatre organismes extraparlementaires, soit une baisse de près de 19 % par rapport à aujourd'hui. Enfin, je me félicite que la commission des lois ait souhaité que les parlementaires soient plus étroitement associés aux travaux de la commission départementale de la coopération intercommunale- la fameuse CDCI -, sans voix délibérative toutefois, de sorte à préserver l'autonomie et l'indépendance des élus locaux.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, une analyse rapide pourrait faire apparaître le présent texte comme la simple conséquence des lois pour la confiance dans la vie politique, notamment l'article 13 de la loi organique, alors qu'il est aussi l'aboutissement d'un travail de longue haleine, engagé par le groupe chargé de réfléchir sur les méthodes de travail du Sénat en 2014, loin des polémiques et de la démagogie qui parasitent trop souvent les débats sur le fonctionnement de nos institutions. Au-delà de l'harmonisation et des clarifications auxquelles il procède, ce texte pose incidemment la question de l'organisation du travail et des missions des parlementaires, réflexion d'autant plus utile que nous examinerons prochainement une réforme de la Constitution qui prévoit des dispositions relatives à la procédure législative et aux droits du Parlement. Dans cette attente, la présente proposition de loi a entamé un recensement et une évaluation de tous les organismes extérieurs au sein desquels siègent des parlementaires et procède à une simplification et à des rationalisations qui sont bienvenues. Ce patient travail a été réalisé en collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat, comme en témoigne le dépôt concomitant de deux propositions de loi identiques.

législative et politique des parlementaires, mais aussi alimenter les parlementaires qui y siègent et éclairer leur travail législatif et de contrôle. J'attire votre attention sur les implications de la présence de députés et de sénateurs au sein des OEP. Les consultations menées par M. le rapporteur indiquent que cette présence est particulièrement appréciée, car elle assoit la légitimité de leurs décisions. Une question se pose toutefois, lorsque des parlementaires siégeant au sein d'un OEP n'en partagent pas les orientations et ne tiennent plus à lui apporter leur caution. Je n'en fais pas mystère, c'est une situation que j'ai vécue au sein de l'Observatoire de la laïcité où, compte tenu de sa composition, la voix des parlementaires, réduits au rang de spectateurs impuissants, Il importe aussi de veiller à un bon équilibre, s'agissant du travail et du temps que les parlementaires sont en mesure de consacrer à ces organismes. La diminution prévue du nombre de députés et de sénateurs donne plus d'acuité encore à cette préoccupation.

ne suscite pas d'opposition parmi les sénateurs de notre groupe. Nous regrettons en revanche que nous ne soyons pas parvenus à un accord sur la rédaction de l'article 1 et la notion de représentation des groupes politiques au sein des organismes. La rédaction issue des travaux de la commission des lois apporte toutefois une amélioration par rapport à celle de l'Assemblée nationale, notre groupe étant attaché au respect du pluralisme, et notamment à la représentation des groupes d'opposition ou minoritaires.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Ce texte a fait l'objet d'un dépôt parallèle par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Notre Haute Assemblée, en particulier, s'était déjà intéressée à cette question à l'occasion de la mission conduite en 2015 par le groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, dont nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard étaient les rapporteurs. De manière plus générale, la proposition de loi reflète une préoccupation commune : favoriser l'efficacité de l'information parlementaire et la clarté de la séparation des pouvoirs. séparation des pouvoirs. En premier lieu, les organismes extraparlementaires remplissent un rôle important dans la bonne information du Parlement, en ouvrant une fenêtre sur l'expertise de terrain, dont nous avons indéniablement besoin pour contrôler correctement l'action gouvernementale. clarté dans la séparation des pouvoirs, parce que le paysage des OEP est extrêmement diversifié, allant des comités de suivi instaurés par une loi idoine au conseil de surveillance d'un organisme aussi vénérable que la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'ici, les nominations des parlementaires au sein de ces institutions étaient prévues aussi bien par la loi que par décret, sans qu'aucune règle n'y préside. Dès lors, le flou normatif qui qui régnait sur les nominations de parlementaires était préjudiciable à la bonne séparation des pouvoirs exécutif et législatif. Dans cette optique, la présente proposition de loi tire les conséquences de la récente loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment de son article 13 qui dispose qu'un parlementaire ne peut désormais être désigné, en tant que tel, dans un organisme extraparlementaire

d'abord, en généralisant l'application du principe de parité dans les procédures de nomination, puis en prévoyant que ces nominations refléteront la configuration politique des deux assemblées. Enfin, d'autres dispositions fixent la marche à suivre dans le cas où un parlementaire présidant l'un de ces organismes Dans un second temps, cette proposition de loi procède à un important effort de rationalisation et de simplification du paysage des organismes existants, effort qui résulte des travaux des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat.

et reflètent la grande diversité de cette source d'information pour le Parlement : on trouve, par exemple, le Conseil national de l'habitat, l'Institut des hautes études de défense nationale ou encore l'Observatoire de la laïcité. Ensuite, le même effort conduit à donner une base légale à la présence de députés et de sénateurs au sein d'organismes créés par des lois qui n'avaient pas explicitement prévu la présence de parlementaires en leur sein. Là encore, plus d'une trentaine d'organismes sont concernés, dont le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. En somme, la présence des sénateurs et des députés au sein de ces deux types d'organismes sera régularisée, apportant un surcroît bienvenu de clarté dans cet aspect de la séparation des pouvoirs. Enfin, l'effort de simplification se traduit par la suppression de la présence de droit de parlementaires au sein de certains organismes peu actifs ou au sein desquels leur présence paraît peu justifiée. Cette suppression passe évidemment par le retrait explicite des dispositions prévoyant leur présence, mais aussi par la simple omission de certains organismes. La présence des députés et sénateurs au sein de ces derniers demeurera donc dépourvue de base légale et devra cesser.

au terme de nombreuses concertations et réflexions préalables. La commission des lois a également inclus d'autres organismes dans cet effort de rationalisation. En outre, elle a souhaité la présence de parlementaires dans des institutions où ils étaient jusqu'ici absents, comme le Conseil national de l'air ou le La présence des parlementaires au sein des commissions départementales de la coopération intercommunale, qui a fait l'objet d'un débat en commission, a été maintenue. Elle est le fruit d'une rédaction de compromis, comme l'a rappelé Enfin, la commission des lois a également choisi d'avancer la date d'entrée en vigueur de la loi : initialement prévue en 2022, celle-ci a été ramenée au lendemain de sa publication. En somme, cette proposition de loi est le symbole d'un travail parlementaire productif et moderne

correctement le Gouvernement. Ce cheminement illustre bien l'efficacité de nos institutions et du bicamérisme français, en dépit des critiques qui leur sont parfois adressées. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi qui, à ses yeux, va dans le bon sens. La parole

et le législatif. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d'honneur de Mme Aliona Shkroum, coprésidente du groupe d'amitié Ukraine-France de la Rada d'Ukraine. Notre collègue accompagne le président de la Rada d'Ukraine, qui était en déplacement à Paris et a été reçu en audience hier par le président du Sénat. Cette visite témoigne de l'intensité de la coopération parlementaire, qui s'est nouée ces dernières années entre nos deux assemblées. Malgré le conflit qui sévit encore à l'est de l'Ukraine, des réformes d'ampleur sont conduites dans ce pays à travers les différents secteurs de la vie publique, notamment en faveur de la décentralisation. L'Ukraine a choisi de prendre pour modèle la décentralisation conduite par notre pays depuis une quarantaine d'années. C'est pourquoi, dès 2015, le président Gérard Larcher a souhaité que l'expérience acquise par le Sénat en ce domaine soit mise à la disposition de nos collègues ukrainiens. le Sénat a accueilli plusieurs délégations de parlementaires et de fonctionnaires pour accompagner l'Ukraine dans cette réforme de la démocratie locale. Le groupe d'amitié France - Ukraine du Sénat, présidé par notre collègue Hervé Maurey, que je salue également, prend toute sa part à cet effort en vue de pérenniser des échanges de travail fructueux. Je formule le voeu que cette visite affermisse encore les liens entre nos deux parlements et, à travers eux, nos deux nations. Soyez, madame la présidente, la bienvenue au Sénat français

côté positif, on notera l'adjonction de parlementaires dans des organismes où ils n'étaient pas présents, ainsi que l'institution de la règle de la parité dans le processus de nomination par les assemblées. À l'heure de la simplification, j'avoue cependant que le soin mis à préciser le détail de ces règles a suscité mon admiration

J'en conviens pour les nominations dans des organes à vocation technique, sans portée politique ; pour les autres, tels le Comité des finances locales, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ou le conseil d'administration de l'Agence française de développement, il me semble qu'il en va tout autrement. Certes, les majorités auront toujours le dernier mot, mais les groupes minoritaires pouvaient au moins s'exprimer lors des débats qui accompagnaient généralement ces nominations. Je m'interroge

Comme on le voit, ce texte qui embrasse beaucoup- on parle de cent quatorze organismes -étreint finalement peu. Je confirme ce que j'ai dit en commission : le groupe CRCE s'abstiendra sur ce texte.

quatre présidents de groupe de l'Assemblée nationale et déposée en termes identiques par le président du Sénat, la troisième vice-présidente et les présidents de nos huit commissions. De plus, l'examen de ce texte a été, une fois encore,

Je salue, dans cette optique, le travail de notre rapporteur, Loïc Hervé, qui a mené les débats de manière sereine et qui a permis d'améliorer substantiellement le texte qui nous était proposé. Sur le fond, ensuite, cette proposition de loi a trait au bon fonctionnement et à l'organisation des instances extérieures aux assemblées. Ces organismes extraparlementaires, parce qu'ils sont souvent vecteurs de débats, d'expertises et d'idées, font partie des outils au service de l'activité démocratique de notre pays. La présence de parlementaires au sein de ces organismes est souvent nécessaire : elle participe indirectement

cents organismes extraparlementaires recensés sont toutefois extrêmement différents, tant par leur statut que par leur niveau d'activité, composition ou domaine d'expertise. Il est donc nécessaire d'harmoniser ce système pour le simplifier. Adoptée en septembre dernier, la loi organique pour la confiance dans la vie politique a modifié le code électoral, afin de prévoir qu'un sénateur « ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ». L'objectif de cette réforme était double : il s'agissait, d'une part, de limiter la multiplication des organismes et, d'autre part, de respecter la séparation des pouvoirs, laquelle exige que la présence d'un parlementaire soit prévue par la loi, et non par un simple décret. En effet, depuis 2014, soixante nouveaux organismes ont été créés Il est évident que c'est trop. Et que ce soit par la loi ou par des actes réglementaires, un peu plus de deux cents organismes prévoient la présence des parlementaires. C'est encore une fois beaucoup trop. Aussi est-il nécessaire de limiter la prolifération de ces instances et de clarifier les règles régissant la présence des parlementaires afin de de rationaliser leur fonctionnement. Personnellement, au cours de mes précédents mandats au Sénat, j'ai été nommé dans des organismes qui ne se sont jamais

Je pense notamment à la Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice- j'ai attendu pendant des années d'y être convié ! -ou encore à la Commission consultative pour la production de carburants de substitution,

Parce qu'il est nécessaire de passer d'une égalité de principe à une égalité réelle, ce texte est important. Dans cette perspective, la proposition de loi mentionne explicitement l'objectif d'un partage réel des postes et des responsabilités entre les femmes et les hommes. Très bien ! Le caractère paritaire est ainsi consacré dans toutes les procédures de nomination et de remplacement des parlementaires au sein des organismes extérieurs au Parlement. plus que la simplification et la précision que ce texte apporte, son enjeu principal est de distinguer ceux des organismes qui seront ou non élevés au rang législatif de ceux qui seront supprimés. À ce propos, les débats en commission ont porté sur l'opportunité de viser explicitement tel ou tel organisme. C'est ainsi que la commission des lois a décidé de supprimer du champ de la proposition de loi la Commission de concertation du commerce, la Commission nationale des services ou encore le Conseil national des professions du spectacle. De même, des organismes jugés obsolètes ou trop peu efficaces sont supprimés, tels que le comité chargé de suivre un rapport du Gouvernement sur la protection des mineurs à l'égard de contenus audiovisuels susceptibles de leur nuire

À l'inverse, certains organismes ont été ajoutés, parce qu'ils revêtent une importance particulière et que leur absence dans un tel texte constituait une erreur. C'est le cas, par exemple, du Conseil national de l'air. Je n'ai pas cité ici toutes les modifications faites par la commission des lois sur la proposition de son rapporteur,

discuter de la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Ce texte a fait

de révision de la carte des intercommunalités. La première a été mise en oeuvre au 1 janvier 2014, la seconde au 1 janvier 2017. Nos collectivités ont besoin de stabilité

pour la création d'une intercommunalité. Le gouvernement de l'époque disait 20 000 ; nous disions 10 000 ; nous nous sommes entendus sur 15 000. Mais nous n'avons jamais discuté de la population maximale qu'il serait réaliste de prévoir dans les intercommunalités rurales, si bien que les préfets, parfaitement légalement du reste, ont pu dans certains départements modeler la carte des intercommunalités, imposant souvent leur décision par voie d'autorité, certes après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et vote des conseils municipaux. Se sont ainsi constituées d'énormes intercommunalités rurales, dont certaines ont d'ailleurs pris le nom- c'est assez piquant -de « communauté d'agglomération », alors qu'elles sont entièrement composées de territoires ruraux, avec, parfois, de petites villes

de loi vise à combler ce vide et organiser cet espace, en donnant une réalité plus forte aux pôles territoriaux qu'un certain nombre d'intercommunalités, d'ailleurs, ont eu l'intelligence de mettre en place, mais sans pouvoir, sur

des élus. Cela n'empêchera pas la commission départementale de la coopération intercommunale de continuer à réfléchir aux aménagements, notamment pour les syndicats intercommunaux qui subsisteraient encore après ces deux vagues de révision de la carte, de délibérer et d'avoir naturellement ses propres idées.

soient élargies, par délégation de l'État, dans les domaines de la politique de l'emploi et de l'enseignement supérieur. Telle est, mes chers collègues, l'économie générale de cette proposition de loi, qui va maintenant faire l'objet de nos débats.

mûrie à l'écoute des élus locaux, est donc très simple : améliorer sans perdre de temps ce qui doit l'être et, surtout, supprimer les entraves,

Mais quel législateur serions-nous si nous restions indifférents à des dysfonctionnements manifestes, à des rigidités excessives, dont une écrasante majorité d'acteurs locaux dénoncent les méfaits ?

qui traversent parfois des difficultés lourdes, notamment dans les secteurs ruraux ou périurbains, des raisons de croire et d'espérer. Ce sera, Ce sera, en somme, « l'agence du quotidien » et elle pourra réellement changer la donne pour nos concitoyens qui vivent en marge des territoires métropolitains.

J'en viens rapidement à la question, cruciale, de la revitalisation de l'échelon communal et à l'assouplissement des conditions de la coopération intercommunale. Non, je le dis avec force, la commune- le bloc communal -n'est pas une entité recroquevillée sur elle-même, dépassée par son époque. Les organisations, les schémas, les regroupements se font et se défont au gré des modes, mais les communautés humaines demeurent. C'est au sein de la commune que se tisse le lien social le plus solide, le plus pérenne. C'est dans les villes et les villages que les femmes et les hommes font l'apprentissage de la solidarité, de la capacité à mener des projets communs, de la prise de responsabilités associatives ou électives, mais aussi des difficultés, bref, des difficultés, bref, du fait qu'en plus d'être des habitants, ils peuvent investir pleinement leur condition de citoyen. Si elle demeure favorable au mouvement de création des communes nouvelles, la commission des lois

plus exhaustif et approfondi à l'occasion de la discussion prochaine de la proposition de loi présentée par notre collègue Françoise Gatel. S'agissant de l'intercommunalité, lois a souhaité concilier deux principes essentiels. Le premier consiste à ne pas défaire les cartes intercommunales qui viennent d'être redessinées et que les communes tentent,

à celles qui connaissent les situations les plus complexes du fait de mariages forcés souvent unanimement reconnus, y compris au sein des EPCI, de s'en affranchir, tout en offrant aux intercommunalités, bien évidemment de manière encadrée, la capacité de surmonter ces blocages. Nous avons donc apporté certains assouplissements aux conditions actuelles de la coopération intercommunale, en octroyant à un groupe de communes contiguës le droit de se retirer d'un EPCI pour constituer un nouvel établissement. Mes chers collègues, en 2018, nous croyons encore- même plus que jamais -à la décentralisation, non pas comme un totem ou parce qu'elle serait inscrite dans notre Constitution, mais parce que tous, ici, nous avons constaté que les bonnes décisions sont celles qui coïncident avec la réalité.

le président Philippe Bas y faisait référence s'agissant des régions, nous nous plaçons délibérément à contre-courant du mouvement de recentralisation de la formation professionnelle engagé par le Gouvernement. Avec cette proposition de loi, Avec cette proposition de loi, nous voulons donner à la région les moyens de coordonner les acteurs publics de l'emploi et l'associer plus étroitement à la gouvernance de Pôle emploi. De plus, la commission des lois a prévu divers mécanismes pour renforcer le rôle des régions dans le pilotage national de la politique d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que dans la gouvernance des établissements. Nous avons pu avoir des débats antagonistes, ici même, au moment de la création des grandes régions. Je ne prétends surtout pas rouvrir ce débat aujourd'hui. Mais dès lors que cet outil existe, utilisons-le

nous assistons aujourd'hui, dans notre pays, à une baisse très sensible des vocations et de l'engagement civique. Ce désintérêt pour l'exercice des mandats locaux est un phénomène

prochainement des propositions. Sans préjuger de ces conclusions, nous avons déjà souhaité apporter des réponses à deux motifs de préoccupation, régulièrement avancés par les élus : la difficulté de concilier leur mandat avec leur vie professionnelle et les risques juridiques qu'ils courent. La commission des lois a donc adopté des dispositions visant à renforcer le statut des élus locaux, en facilitant la conciliation de l'exercice d'un mandat avec une profession salariée ou en réduisant les risques juridiques pesant notre commission a approuvé diverses mesures destinées à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales. Ces mesures concernent notamment la délégation partielle de compétences, ainsi que d'autres dispositions techniques, techniques, circonstancielles, mais là aussi, très attendues par l'ensemble des élus. Certes, je ne prétends pas émouvoir outre mesure cet hémicycle en citant la faculté, que nous avons introduite, de percevoir un droit de timbre pour l'instruction des autorisations

tant que faire se peut, la tâche de celles et ceux qui, quotidiennement et au prix de lourds sacrifices, mettent leur énergie au service de nos concitoyens. Nous le devons

entend prouver dans les débats à venir qu'il joue un rôle indispensable dans nos institutions, c'est en légiférant, ici et maintenant, au service de nos territoires. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a examiné au fond, sur délégation de la commission des lois, les sept articles du titre I de la proposition de loi dont nous avons à connaître aujourd'hui. Ces articles ont pour objet de créer une agence nationale pour la cohésion des territoires. La commission considère que cette proposition arrive au bon moment, alors que le Président du Sénat et de nombreux élus souhaitent la réalisation de ce projet depuis plus d'un an et que le Président de la République a annoncé la création d'une telle agence lors de la réunion de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017.

Je rappelle, à cet égard, que parmi les vingt-six propositions que nous avons formulées en 2017, avec le président Hervé Maurey, dans notre rapport d'information consacré à l'aménagement du territoire, figurait déjà l'idée de créer un guichet unique au service des territoires ruraux et périurbains pour répondre à leurs besoins en ingénierie et en conseil. Je salue donc l'initiative de nos collègues, qui montre la détermination du Sénat à inventer des solutions pour ces territoires. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable partage le parti pris des auteurs de la proposition de loi de s'inspirer, pour constituer la nouvelle

Nous avons plus que jamais besoin d'une politique volontariste d'aménagement du territoire et de rééquilibrage territorial face à une polarisation croissante entre les métropoles dynamiques et les petites villes, les campagnes et les bourgs, qui constituent les territoires ruraux et périurbains. La commission a apporté plusieurs modifications au texte pour assurer la prise en compte du développement durable dans les actions menées par l'Agence et préciser ses modalités de fonctionnement afin de lui donner une assise juridique solide et cohérente avec ses missions. Je tiens également à saluer le travail réalisé par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin dans leur proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Nos réflexions convergent et l'agence de revitalisation qu'ils proposent aura certainement vocation à s'intégrer à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires.

et fédérer les énergies et à rationaliser l'intervention de l'État dans la politique de cohésion. Nous ne voulons pas créer un nouveau guichet J'attire votre attention, madame la ministre, sur la nécessité de prendre, sans délai, les mesures visant à répondre à une demande forte d'accompagnement des territoires et de soutien en ingénierie technique et financière pour favoriser leur développement. Je remarque qu'il serait sans doute peu opportun que cette nouvelle agence soit créée par décret, car cela empêcherait la représentation nationale d'apporter son éclairage sur les besoins des territoires, auxquels elle sera censée répondre, et de contribuer à la définition de la meilleure structure organisationnelle possible pour mener à bien les missions de l'Agence. Pourriez-vous, madame la ministre, nous donner des précisions supplémentaires sur ce front et, au-delà, sur le calendrier de création de l'Agence ?

et à la vitalité de la démocratie locale qu'il nous est donné d'examiner aujourd'hui est une excellente occasion de débattre d'un sujet très structurant : la cohésion des territoires. Collectivement, État, collectivités territoriales, mais aussi acteurs semi-publics et privés, nous devons répondre au défi des fractures territoriales. Nous partageons les préoccupations des auteurs de cette proposition de loi, mais nous considérons que seule une politique volontariste d'ensemble en matière de cohésion des territoires permettra de répondre au besoin d'équilibre territorial. Nous souhaitons que chaque Français, qu'il naisse ou grandisse au coeur d'une grande ville, dans un quartier en politique de la ville, dans une commune périurbaine ou d'outre-mer ou dans un village de montagne, puisse avoir les mêmes chances. Les oppositions entre l'urbain et le rural, les métropoles et la France dite périphérique, doivent être dépassées au profit d'une vision dynamique et solidaire. Tous les territoires représentent un potentiel de développement pour leurs habitants et le pays tout entier. Face à la perception grandissante, au cours des vingt dernières années, d'une lente dégradation des conditions de vie et d'un déclassement que l'application uniforme de mesures nationales pourrait accentuer, la politique des territoires doit rechercher des mesures volontaristes dans leur ambition, concrètes dans leurs effets et adaptées à chaque territoire dans leur mise en oeuvre. Pour ce faire, nous souhaitons que des leviers soient activés. d'abord, au levier de la transition numérique, régulièrement débattu dans cet hémicycle, pour lutter contre l'exclusion d'une partie des Français. L'outil numérique est un atout pour concilier modernisation et accès aux services publics essentiels

également développer la différenciation entre les modes d'intervention. Plutôt que d'imposer partout les mêmes compétences ou modalités de mise en oeuvre de ces dernières, le Gouvernement souhaite adapter l'élaboration et l'application des réformes à la diversité des enjeux locaux. C'est ainsi que le dispositif Action coeur de ville se déploie dans l'Hexagone et en outre-mer. C'est également- nous y reviendrons, bien sûr -le sens de l'inscription dans la Constitution du principe de différenciation, qui pourrait permettre à deux collectivités d'une même catégorie d'exercer des compétences différentes ou de les exercer d'une manière différente.

les auditions nécessaires à la réalisation de sa mission ; il remettra son rapport de préfiguration dans les tout prochains jours. Le Gouvernement a fixé une ligne directrice

qui partent des propositions politiques des élus. Nous aussi ! Nous souhaitons tout à la fois que cette agence soit un guichet unique, un outil de financement et un apport en ingénierie et en conseil.

Enfin, il convient de faire évoluer nos façons de travailler. Le Gouvernement a souhaité engager, avec les collectivités territoriales, un dialogue et une relation de confiance dans le cadre de la Conférence nationale des territoires,

Dans le cadre de la Conférence nationale des territoires a été ouvert un chantier relatif aux conditions d'amélioration de l'exercice des mandats locaux. En outre, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat

Il me semble primordial de respecter cette méthode, et donc de renvoyer l'examen des articles 19 et 20 à un futur véhicule législatif plus global et mieux partagé. Notre modèle français, attaché à l'égalité et à l'équilibre, est marqué depuis une trentaine d'années par plusieurs transformations majeures, que les précédents orateurs ont aux conséquences des révolutions économiques successives- agricole, industrielle et numérique -dans les territoires, à l'essor des métropoles, qui sont devenues des moteurs de la croissance économique, pour elles-mêmes, mais aussi, parfois, pour les territoires avoisinants, quand elles jouent le jeu de la solidarité, ou à l'évolution constante des rôles respectifs de l'État et des collectivités territoriales dans la gestion du développement et des solidarités. Il est vrai qu'en matière institutionnelle, plusieurs réformes successives ont profondément fait évoluer la répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités territoriales, afin de rendre l'action publique la plus claire, la plus lisible et, bien sûr, la plus efficace possible. Depuis la loi Chevènement de 1999 sous tous les gouvernements, quelle que soit la majorité au pouvoir, l'intercommunalité s'est développée et transformée. Mais c'était de manière volontaire ! Sur le plan institutionnel, dite RCT, a rendu obligatoire le regroupement des communes en EPCI à fiscalité propre.

Les articles 12 à 16 visent à élargir le champ d'intervention des départements. De ce fait, ils contreviennent à la répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités territoriales issue de la loi NOTRe, qui a notamment mis fin à la clause de compétence générale pour les régions et les départements. À nos yeux, la clause de compétence générale doit être conservée pour les communes, premier échelon de proximité, mais la répartition des compétences entre les autres niveaux de collectivités doit rester stable et lisible. Les articles 17 et 18 visent à spécifier le rôle des régions en matière de politique de l'emploi et de formation supérieure.

Enfin, les articles 20, 21 et 22, ainsi que ceux introduits en commission, paraissent de nature à alourdir le fonctionnement des EPCI plutôt qu'à les rendre souples et adaptables.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner une proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale. L'empressement de ses auteurs témoigne de la détermination du Sénat à agir au service des territoires. C'est évidemment tout à notre honneur Cet empressement semble dicté par la nécessité d'opérer certains ajustements aux récentes réformes territoriales, la loi du 7 août 2015 dite NOTRe en tête. Naturellement, ce travail doit être mené sans galvauder l'architecture de l'organisation territoriale de la République et l'esprit qui en émane. Si des ajustements ponctuels sont inévitables- ainsi, de concert avec Mme la ministre, nous venons d'améliorer l'exercice des compétences eau et assainissement sans bouleverser les territoires -, ce texte est de nature à fragiliser les arrangements qui viennent d'être trouvés. Comment ne pas s'étonner de voir cette initiative sénatoriale présentée comme un texte d'ajustement ? Tel n'est sans doute pas

Entendons-nous bien : nous allons débattre de l'opportunité de créer une agence nationale pour la cohésion des territoires, en principe dédiée aux besoins d'ingénierie et d'accompagnement des territoires ruraux et périurbains

étonnant : celui de ramasser au sein d'un même véhicule législatif des dispositifs d'affichage-

les élus, ne revenons pas prématurément et de manière incomplète et instable sur les textes qui ont institué les recompositions territoriales. Faisons confiance aux élus locaux ! Et puis, convenons-en, cet assemblage de dispositions,

interpeller ! Ce texte vise à créer une agence nationale pour la cohésion des territoires, à apporter plusieurs assouplissements aux conditions actuelles de la coopération intercommunale, à consolider les compétences départementales en matière de solidarité territoriale, à régionaliser les politiques de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à renforcer le statut des élus locaux. Or nous ressentons, chez nos élus, une grande lassitude face aux modifications successives de la

Eh bien, faisons-le et évitons des textes partiels, alors même que des travaux de fond sont engagés par ailleurs. L'aspect véritablement novateur du texte, ce sur quoi il convient de porter notre attention, réside dans la création de l'Agence il paraît prématuré de débattre de son champ d'intervention territorial, des missions qui lui seront assignées et de l'épineuse question de son statut juridique. Le préfigurateur rendra ses conclusions dans les prochains jours et les arbitrages seront ensuite attendus. Fixer les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette structure, sans même attendre l'aboutissement du travail de préfiguration, n'a sans doute pas de sens. En revanche, divers sujets, comme la responsabilité, la formation, l'apprentissage, l'emploi, le statut des élus simplification de la vie et de l'organisation des territoires, méritent évidemment, chacun, un texte approfondi, global, donnant durablement de la visibilité et de la stabilité. Ces travaux utiles existent.

Enfin, je tiens à insister sur un dernier point. Le rythme du travail gouvernemental est une chose ; le rythme du travail du Sénat en est une autre. Nous vivons sous un régime de séparation des pouvoirs. Nous ne sommes pas tenus d'attendre que le travail gouvernemental soit arrivé à maturité, surtout quand il est lent- et c'est le cas en l'occurrence. Un an ! Je rappelle que le Président de la République s'est exprimé, après le président du Sénat, lors de la réunion de la Conférence des territoires du 17 juillet dernier et l'on en est encore au stade de la mission de préfiguration Je n'en porte pas grief au titulaire de cette mission ; il a lui-même été désigné tardivement. Mais enfin, monsieur de Belenet, vous nous demandez d'attendre que le commissaire général à l'égalité des territoires ait

selon laquelle le Parlement ne pourrait jamais débattre et se prononcer par des textes de loi sans que le Gouvernement l'ait saisi.

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

l', bateau affrété par SOS Méditerranée, a recueilli le 9 juin 629 personnes, dont 123 enfants mineurs isolés

Ma question est simple, monsieur le Premier ministre : la France est-elle prête à respecter son devoir humanitaire, celui que le président de la République avait exprimé avec Mme Merkel, le 23 juin 2017 ?

auraient dû permettre à ce bateau d'être accueilli dans le port le plus proche, soit à Malte, soit en Italie. Le gouvernement italien n'a pas souhaité le faire. C'est une contradiction au regard des règles internationales et, d'une certaine manière, c'est une rupture par rapport à l'action que menait le précédent ministre de l'intérieur italien, lequel avait réussi à à contenir les passeurs envoyant parfois à la mort à travers la Méditerranée des dizaines, voire des centaines, de milliers de migrants. Nous devons reprendre les règles normales et faire en sorte qu'il y ait cette responsabilité pour les pays qui doivent accueillir. J'ai parlé ce matin au téléphone avec le ministre de l'intérieur espagnol et je l'ai assuré de la solidarité de la France. Nous nous sommes longuement entretenus afin de définir une position commune européenne et nous serons, avec le Président de la République, à Berlin, mardi prochain, pour dire ce que devraient être les règles d'une coopération européenne en matière de migration. au téléphone avec le ministre italien de l'intérieur, à qui j'ai rappelé qu'il convenait d'avoir des règles européennes communes et, en particulier, de respecter les accords de coopération qui existent entre la France et l'Italie.

Nous devons ainsi faire preuve de solidarité quand un de nos voisins fait face à des arrivées massives de réfugiés ou de migrants. » Non ! L'Italie est confrontée à ce phénomène, et on le sait depuis longtemps. L'article 13 du règlement de Dublin oblige censément l'Italie à instruire les demandes d'asile de toutes ces personnes. Le Président de la République lui-même a dit, il y a un an, que nous devions trouver une réponse, mais vous vous évertuez encore à faire appliquer ce règlement de Dublin qui ne tient pas

Le Président Trump, qui avait déjà refusé de signer la partie du communiqué conjoint sur le climat, a retiré entièrement la signature des États-Unis, dans l'avion qui l'emmenait vers Singapour. Face à ce caprice, votre homologue allemand a déclaré : « En quelques secondes, vous pouvez détruire la confiance en 280 caractères sur Twitter.

Comment faire confiance à un allié qui déchire ses engagements sur l'Iran et menace les entreprises européennes de représailles ? Comment faire confiance à un allié qui remet en question le principe même de l'Alliance atlantique, en affirmant qu'elle lui coûte trop cher ? Pendant ce temps, Vladimir Poutine, qui rencontrait ses homologues chinois et iranien, avait beau jeu d'ironiser sur le « babillage inventif » des pays du G7. Madame la ministre, face à l'imprévisible M. Trump, il est temps que l'Europe devienne enfin une puissance capable de négocier en position de force. Il est temps que l'Europe relève le défi de l'unité et de la cohésion pour parler d'une seule voix face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Ma question est la suivante : quelles initiatives la France compte-t-elle prendre pour tirer les conséquences de l'échec du G7 de Charlevoix et pour, enfin, construire une Europe indépendante, souveraine et puissante ? La parole

vous avez raison, le sommet du G7 s'est mal terminé et nous le regrettons. Un travail important avait été accompli, un accord était intervenu sur un texte ; il n'est jamais bon de revenir sur un accord signé. Je voudrais partager avec vous deux convictions. La première, c'est que nous avons besoin d'un cadre multilatéral efficace pour traiter les enjeux globaux, qu'il s'agisse du commerce, du climat, de la santé ou du terrorisme. Nous en avons besoin, comme les États-Unis en ont besoin. En l'absence d'un tel cadre, c'est la loi de la jungle qui l'emporte et personne n'est gagnant. Ma seconde conviction, c'est que les États-Unis sont pour nous un partenaire et un allié,

Avec l'administration du Président Trump, des divergences, nous en avons : sur le commerce, sur l'accord nucléaire avec l'Iran, sur l'accord de Paris, sur Jérusalem, nous ne sommes pas d'accord, et nous le disons.

nos intérêts propres. L'alliance n'interdit pas, bien au contraire, de faire valoir nos intérêts, à titre national et à titre européen. C'est ce que nous faisons en décidant de mesures de rétorsion et de mesures de sauvegarde face

Nous avons besoin d'une Europe plus unie, plus forte et plus souveraine. C'est ce que le Président de la République a proposé et c'est à cela que nous travaillons. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour le groupe Les Républicains. Monsieur

Cet homme a naguère posé avec un tee-shirt portant la mention « Jihad » en lettres d'or sur fond noir. Pour qu'il soit bien clair que le jihad dont il était question n'était pas uniquement une réforme personnelle et morale, comme le veulent les tenants de la, le « J » initial y était figuré par un sabre,

C'est cette période qui vit l'abrogation des versets coraniques favorables à la liberté religieuse et à la coexistence pacifique avec les juifs et les chrétiens, par d'autres versets coraniques invitant à massacrer et à réduire en esclavage les non-musulmans. C'était au VII siècle Aujourd'hui, au XXI siècle, un examen rapide sur internet permet de retrouver bien des paroles de ce rappeur. Il y fait l'éloge de la polygamie, invite à crucifier les « laïcards » ou se propose d'émettre des sur les gens qui ne lui reviennent pas.

serais pourtant curieux de savoir quel contexte justifie des appels au meurtre ! On peut présenter toutes les arguties que l'on voudra, la réalité, dans sa cruelle simplicité, c'est que le théâtre de l'une des tueries les plus sanglantes jamais perpétrées sur notre sol va recevoir un apologiste du jihad et de l'islam radical

les sénateurs, mais ce n'était pas le cas la semaine dernière, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la programmation du Bataclan et sur le fait que le rappeur que vous avez mentionné s'y produise.

ceux qui aujourd'hui le font vivre et l'ont remonté ont choisi librement la programmation que vous critiquez. Monsieur le sénateur, c'est peut-être honteux pour vous, mais ils ont choisi cette programmation.

la loi. S'agissant d'un concert, s'agissant du choix libre effectué par une salle de sa programmation, la loi est très simple.

poursuivre ! Mesdames, messieurs les sénateurs, j'essaie de m'exprimer calmement sur un sujet qui vous touche autant que moi, et j'essaie de rappeler, car cela ne me semble pas déplacé

Nous respecterons donc scrupuleusement et la liberté d'expression et la loi. C'est la ligne du Gouvernement, ... Je n'ai pas de mots ! ... et nous la tiendrons en

qui ont trouvé la mort ou qui étaient présents ce soir-là.

c'est une élue rurale qui s'exprime devant vous, une élue qui ne supporte plus l'abandon du monde paysan. Le constat est cinglant : nos agriculteurs sont à bout ! Hier encore, alors que je visitais des exploitations dans le département de l'Essonne, ces derniers m'indiquaient qu'ils n'en pouvaient plus. Nous pouvons être fiers de leur engagement au service de la France, nous pouvons être fiers de la ruralité, je tiens à le souligner. Toutefois, nos agriculteurs ne veulent plus de discours, ils attendent des engagements forts.

En Île-de-France, plus d'un agriculteur sur deux produit du colza. C'est donc toute une filière qui est menacée. La production nationale de colza pourrait enregistrer une perte de surface de 400 000 hectares. Cela ne sera pas sans conséquence sur la production de tourteaux, destinée à l'alimentation des animaux. L'incompréhension est mêlée à un sentiment d'injustice. Sans faire de mauvais esprit, c'est la goutte d'huile qui fait déborder le vase ! Par ailleurs, comment la France va-t-elle justifier cette mesure face aux conséquences écologiques dramatiques qu'elle engendrera en Asie du Sud-Est, sans parler des risques pour la santé ? santé ? Nous ne pouvons pas exiger de nos agriculteurs toujours plus de qualité en leur imposant autant de normes et, dans le même temps, favoriser une concurrence étrangère qui détruirait notre filière d'excellence. Cet effet de ciseaux est insoutenable.

S'agissant de la raffinerie de La Mède, comme vous le savez, Total a décidé en 2015, en accord avec le gouvernement de l'époque, de transformer cette usine en une bioraffinerie de biodiesel. Cette décision a d'abord été prise pour préserver 250 emplois.

créer des débouchés, une filière de recyclage d'huiles usagées, mais aussi de graisses animales, qui sont intégrées à la production à hauteur au moins de 25 %. Total devra également et surtout limiter à 300 000 tonnes sa consommation d'huile de palme. Il est faux de dire que la consommation de ces 300 000 tonnes d'huile de palme va s'ajouter

La parole est à M. Robert Navarro, pour le groupe La République en marche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre chargée des affaires européennes.

À l'avenir, nous ne pourrons compter que sur nos propres forces, c'est une évidence. Dans ce contexte, l'interview accordée le dimanche 3 juin par la chancelière allemande à un grand quotidien, dans lequel elle détaille ses positions sur l'Europe, doit retenir toute notre attention. Mme Merkel répond enfin aux discours ambitieux du Président de la République à Athènes et à la Sorbonne. Nous devons nous en réjouir. Cette interview marque de véritables avancées de la part de l'Allemagne, notamment sur les aspects relatifs Il faut rendre hommage à l'action d'Emmanuel Macron qui, dès mai 2017, a relancé le thème de la défense européenne. Les sceptiques estimaient que c'était une chimère : la preuve est faite, là où il y a une volonté, il y a un chemin L'Europe a besoin d'une force opérationnelle pour monter rapidement une opération de secours au bénéfice de citoyens européens ou une mission d'interposition en Afrique ou en Asie, par exemple. Aussi, je souhaite savoir quelle est l'ambition de la France sur cette question. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer les démarches que vous comptez accomplir pour avancer dans le sens de l'intérêt général de la France et de l'Europe ?

au sud de l'Europe, de la tragédie syrienne à l'instabilité libyenne en passant par les menaces terroristes sur le Sahel, la question de la sécurité de l'Europe se pose de plus en plus.

Ainsi, la coopération structurée permanente a été lancée en décembre de l'année dernière. Dix-sept projets communs, capacitaires et opérationnels, ont déjà été décidés et d'autres sont à venir.

Au-delà même de l'Union européenne à vingt-sept, nous avons proposé un projet d'initiative européenne d'intervention qui permettra d'accentuer notre culture stratégique commune. Nous avons besoin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est l'une des garantes de la sécurité de notre Union.

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le ministre, dans de ce lundi, le directeur de l'UFR de chimie de l'Université Paris-Diderot déplore de devoir refuser des bacheliers de banlieue ayant obtenu d'excellents résultats, au profit de bacheliers parisiens dont les résultats sont, selon lui, moyens, voire médiocres. L'an dernier, sa filière accueillait jusqu'à 40 % d'élèves de banlieue et de province. Cette année, le rectorat a fixé un quota de 3 % dans le cadre de Parcoursup. Selon le directeur, dès la quatorzième place, l'université est obligée de retenir la candidature d'un élève parisien qui plafonne à 8 de moyenne générale, quand un candidat du Val-de-Marne qui a 17 de moyenne se retrouve relégué à la millième place.

Les lycéens de banlieue vont donc se retrouver dans des filières qui ne leur conviennent pas et risquent également d'échouer. Les choses doivent bouger ! À Diderot, les enseignants de la filière biologie ont obtenu que le quota de 3 % de non-Parisiens soit porté à 15 %.

S'agissant de l'académie de Versailles, 34 % des inscrits sur Parcoursup ont obtenu une proposition dans un établissement parisien. Avec APB, ils n'étaient que 21,7

le Val-de-Marne, Paris-XII. Ces universités offrent tout le panel que nous voulons. Si l'on poursuivait jusqu'au bout votre raisonnement, les meilleurs élèves de banlieue iraient au centre de Paris, et il n'y aurait plus de place que pour les moins bons dans les académies limitrophes. Votre raisonnement mènerait à une réelle inégalité, avec des universités de première classe au centre de Paris et de deuxième classe en banlieue. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une approche équilibrée, et c'est ce qui est en train de se passer avec ce que nous avons fait, c'est-à-dire

Ils avaient tous obtenu leur choix pour un BTS, ou même un DUT. C'est le résultat de notre politique, parce que nous avons élargi pour ces lycéens souvent issus de milieux sociaux défavorisés le nombre en DUT et en BTS, c'est-à-dire dans des filières sélectives où ils vont réussir. C'est donc cela, la politique menée et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour en voir les résultats, y compris sur le plan social.

vous appartenez mène une véritable guerre contre les salariés, les retraités, les familles, les jeunes. De la diminution des APL à la hausse de la CSG, vous brisez le caractère solidaire de notre système social au profit d'une vision libérale du chacun pour soi, laissant le champ libre aux appétits des grands groupes privés. C'est précisément dans cette logique que les premières pistes de votre future réforme des retraites évoquent toutes l'objectif de proportionnalité entre les cotisations versées et les pensions versées, sans aucune prise en compte des accidents de la vie et des situations particulières pourtant au fondement du système de protection sociale à la française. Le document de travail du haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, M. Jean-Paul Delevoye, fait peser en ce sens de lourdes menaces sur les pensions de réversion qui permettent aujourd'hui à presque quatre millions de personnes déjà touchées par la suppression de la demi-part fiscale de garder la tête hors de l'eau, et à la solidarité nationale de s'exprimer à l'égard de celles et de ceux qui sont dans l'épreuve. Madame la ministre, il s'agit pourtant du fruit des cotisations de leurs maris le plus souvent, ou de leurs épouses décédées. Ces pensions de réversion permettent par ailleurs de compenser en partie les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Madame la ministre, ma question est simple : quand le Gouvernement cessera-t-il de s'attaquer à ces droits sociaux fondamentaux ?

Devant ce constat, le Président de la République a souhaité proposer aux Français une réforme des retraites visant à rendre notre système plus lisible, plus compréhensible, plus équitable et à redonner confiance à notre jeunesse dans le système des retraites.

concerne les droits contributifs et non contributifs, c'est-à-dire la part de la solidarité dans la réforme des retraites. Aujourd'hui, la part de la solidarité dans les dans les pensions de retraites est de l'ordre de 20 % et il est prévu de maintenir ce ratio. C'est le souhait exprimé par l'ensemble des organisations syndicales. Le document dont vous faites état est un document de travail

Madame la ministre, loin de nous l'idée de faire des procès d'intention. Toutefois, comme on le dit chez nous, chat échaudé craint l'eau froide. Nous avons en effet vu sur différents sujets ce que vous entendiez par concertation- je pense tout particulièrement aux retraités agricoles, à qui vous refusez avec obstination une retraite équivalant une retraite équivalant à 85 % du SMIC. Voilà pour le moins une redistribution qui serait urgente ! La parole

idée : rendre simultanés la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Dans un monde où les carrières professionnelles sont incertaines, on ne peut que louer cet objectif. La mise en oeuvre de cet objectif a été confiée à la haute administration de Bercy, et c'est là que le bât blesse. Un choc de complexification s'est mis en marche. Tout d'abord, en ce qui concerne les crédits d'impôt, les contribuables devront attendre une année avant qu'ils ne produisent leurs effets. Ensuite, le choix entre trois taux, qui nécessitera parfois une régularisation chaque mois, n'est pas de nature à simplifier le dispositif. Enfin et surtout, les entreprises vont devoir se transformer en percepteur. Cela représentera du travail supplémentaire et de nouvelles contraintes en perspective, pour un coût estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Là où il y avait deux acteurs- le contribuable et l'administration fiscale -, demain il y en aura trois. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que les entreprises de notre pays attendent aujourd'hui de la simplification et une baisse de leurs charges ? Enfin, avez-vous pensé à l'incidence de cette réforme sur le pouvoir d'achat des Français ? Vous

Le prélèvement à la source est une bonne idée ; c'est une réforme vertueuse qui permettra d'assurer la contemporanéité de l'impôt payé et des revenus perçus. Aujourd'hui, 90 % des ménages voient leurs revenus varier d'une année sur l'autre, parfois faiblement, parfois de manière plus importante. C'est justement pour prévenir les variations d'impôt sur le revenu qui découlent de cette variation de revenu que nous mettons en place le prélèvement à la source, de manière que l'un et l'autre soient contemporains.

a annoncé que, pour les crédits d'impôt sur les revenus de 2018, les particuliers recevront un acompte au 15 janvier égal à 30 % du crédit d'impôt, et que le solde serait réglé avant l'été de manière qu'ils puissent en bénéficier le plus vite possible. S'agissant du rôle des entreprises, nous veillons nous veillons à simplifier les déclarations au maximum en nous appuyant sur la déclaration sociale nominative, qui est obligatoire, afin de ne pas créer de tâche supplémentaire. Les entreprises se verront

Le prélèvement à la source est une bonne réforme, et le pouvoir d'achat, que vous avez évoqué, ne sera pas touché puisqu'il ne s'agit ni d'une réforme de l'assiette, ni d'une réforme du taux

sur les emplois à domicile ainsi que sur la garde des enfants. Vous aurez peut-être du chômage en plus, vous aurez peut-être du travail au noir, et, surtout, vous ramènerez les femmes à la maison, ce qui n'est pas une bonne chose ! Comme d'habitude, vous faites surtout beaucoup d'agitation,

Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Le Président de la République avait annoncé lors de la COP23, la décision de la France d'en finir avec la production électrique à base de charbon. Cette annonce forte était importante pour crédibiliser notre position dans les négociations climatiques internationales. À la suite de cette annonce, les équipes EDF des centrales thermiques à charbon de Cordemais et du Havre se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour étudier un procédé alternatif à base de biomasse résiduelle et de bois déchets de classe B, et donc sans reproduire l'erreur du mégaprojet de Gardanne de centrale électrique à base de bois coupé, qui était bien évidemment une aberration écologique. Ces expérimentations ont bien avancé. Je laisserai les exploitants donner leurs résultats en détail, mais il apparaît qu'elles sont un succès technique, qu'elles permettent de réduire d'un facteur 40 les émissions de CO2 liées au charbon pour des centrales passant de semi-base à rôle d'appoint, et que la ressource nécessaire est disponible régionalement. Il s'agirait aussi d'une solution d'économie pour les collectivités confrontées à la mise en décharge onéreuse des bois de classe B et des biomasses résiduelles qui encombrent les déchetteries. Le maintien de ces sites apparaît donc comme un outil précieux pour accompagner le développement des énergies renouvelables. De plus, leur préservation offre l'opportunité, dans un futur plus ou moins proche, d'y installer des unités de stockage d'électricité et de production d'hydrogène. Enfin, ces expérimentations peuvent nous permettre d'exporter une technique alternative aux centrales à charbon vers des pays gros producteurs de biomasse, je pense au Kenya, au Nigéria ou à la Côte-d'Ivoire qui envisagent de lancer des investissements charbon. Cet enjeu est peut-être même le plus important. deux questions, madame la secrétaire d'État. Tout d'abord, pouvez-vous nous assurer que le Gouvernement a bien compris tout l'enjeu écologique du maintien d'unités de production électrique de ce type à Cordemais et au Havre ? Ensuite, pouvez-vous nous indiquer un calendrier précis de décision finale de l'État ? La parole

et je vous en remercie. Nous avons spécifiquement lancé une mission interministérielle pour nous aider à déterminer avec précision quelles sont les bonnes façons d'accompagner les territoires autour de chacune des quatre centrales à charbon, l'enjeu étant de faire en sorte que cette transition soit

EDF pour comprendre les contraintes sur le réseau et identifier les possibilités d'évolution de l'outil industriel. EDF étudie par ailleurs la possibilité de faire évoluer les centrales sur place. Concernant plus particulièrement la centrale de Cordemais, des études sont en cours de finalisation. EDF pourra, dans le respect de la contrainte de la fin de l'utilisation du charbon, proposer des pistes soutenables.

vous avez souhaité délocaliser vos conseils des ministres pour être au plus près des Français. L'intention est louable, mais avez-vous entendu, avez-vous compris les Français, qui, dans nos campagnes, dans nos villes, voient leur pouvoir d'achat fragilisé par la succession de taxes et d'impôts que vous leur réservez ? réservez ? Vous avez baissé les allocations familiales, vous avez augmenté la CSG, touchant de plein fouet huit millions de retraités, vous avez maintenu le prélèvement à la source pour janvier prochain, vous avez augmenté le prix des assurances, des mutuelles, du gaz et de l'électricité, du tabac et j'en passe. Vous avez également augmenté le prix des carburants : le prix du pétrole grimpe et en même temps, vous augmentez les taxes sur les hydrocarbures. En un an, le prix de l'essence a augmenté de 6,5 % et le prix du gazole, de 12 %. Depuis 2013, jamais les prix n'ont été aussi élevés. L'usage de la voiture est pourtant indispensable à nos concitoyens en milieu rural pour le travail et pour l'accès aux soins. Les conséquences sont lourdes pour leur mobilité. Dans le « nouveau monde », la vie est chère, trop chère, particulièrement pour les classes moyennes. Nous vivons la saison 2 du choc fiscal, après celui du quinquennat Hollande. Malgré les efforts demandés, plus ou moins justifiés, nos compatriotes ne voient ni l'amélioration de la situation budgétaire de la France, ni la baisse de la dépense publique pourtant nécessaire au redressement de notre pays. Quel est le cap ? Où sont les économies structurelles ? Quelles réponses pouvez-vous nous apporter ?

et dynamique. C'est un acte de foi. Elle vise à rendre aux Français du pouvoir d'achat, à alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, à reporter la fiscalité sur un certain nombre de sujets qui nous tiennent à coeur, comme la transition énergétique. La CSG ! Vous avez noté l'augmentation du prix des carburants. Il est vrai que leur prix a augmenté depuis le début de l'année sous le double effet de la fiscalité et de l'augmentation des cours internationaux du pétrole. Nous ne méconnaissons pas l'impact de cette hausse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais nous prenons des mesures pour protéger les plus vulnérables et pour alléger un certain nombre de charges qui pèsent au jour le jour sur nos concitoyens. Nous baissons les taxes sociales qui pèsent sur les revenus du travail, parce qu'il faut que le travail paye mieux. Nous supprimons progressivement la taxe habitation. Nous apportons grâce au chèque énergie une aide moyenne de 150 euros par an à près de quatre millions de foyers. Nous revalorisons les prestations familiales et l'allocation de solidarité des personnes âgées. En octobre, nous revaloriserons la prime d'activité de 20 euros par mois. Monsieur le sénateur, nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie, qui est celle de la justice, de l'efficacité et de l'équité. La parole Madame la secrétaire d'État, j'entends la communication du Gouvernement, mais les Français vivent dans une autre réalité : augmentations ; diminution du pouvoir d'achat. Un jour, les réalités rattraperont la communication de votre gouvernement.

la culture intensive de l'huile de palme est une des causes majeures de la déforestation, dont l'impact sur le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité a largement été démontré. Apparemment conscient des enjeux, le Gouvernement a affirmé dans l'axe 15 de son plan climat vouloir mettre fin à l'importation en France de produits contribuant à la déforestation. Le même gouvernement a pourtant pris un décret le 16 mai dernier autorisant le groupe Total à importer 300 000 tonnes d'huile de palme par an pour sa raffinerie de La Mède. Quand on sait que plus de 75 % des 900 000 tonnes d'huile de palme consommées dans notre pays sont déjà utilisées comme carburant, on se demande à quoi bon continuer à culpabiliser le consommateur de pâte à tartiner ! Très bien ! Vous me répondrez que ce décret n'émane pas de votre ministère. Certes, mais il illustre de manière criante les incohérences de votre gouvernement. L'arrêté autorisant l'importation de cerises traitées au diméthoate en est un autre exemple. Ce produit phytosanitaire, reconnu dangereux pour la santé, est interdit en France depuis 2016. Peut-être pouvez-vous nous expliquer comment ce produit peut être dangereux quand il est utilisé en France, mais devenir inoffensif lorsqu'il est importé ? La question vaut aussi pour de nombreux produits utilisés en viticulture ou dans la filière fruits et légumes. Dans quinze jours nous entamerons dans cet hémicycle l'examen du projet de loi « agriculture et alimentation ». Nous présenterons alors des amendements permettant de réintroduire de la cohérence entre les pratiques et les substances autorisées sur notre sol et celles qui sont permises pour les produits d'importation. mettrez-vous en cohérence les beaux discours du Gouvernement avec son action ? Serez-vous favorable à notre amendement interdisant l'importation de produits traités avec des substances phytosanitaires interdites en Europe ? La

un climat de dialogue efficace. Depuis plusieurs jours, mon collègue Stéphane Travert, ministre de l'agriculture, est à l'écoute des inquiétudes exprimées par les agriculteurs. Stéphane Travers est actuellement en train de discuter avec la FNSEA et

Il y a beaucoup de Français pour qui c'est la question, il est donc important de le dire ! Depuis le début du quinquennat, la méthode de ce gouvernement c'est le dialogue ; nous en avons d'ailleurs fait la preuve avec les états généraux de l'alimentation.

Je tiens aussi à préciser à nouveau que l'objectif est de substituer une production française à des importations contenant de l'huile de palme. Il est donc faux de dire que la consommation de 300 000 tonnes d'huile de palme à La Mède va s'ajouter à l'utilisation actuelle d'huile de palme dans le secteur des agrocarburants. Nous avons obtenu des avancées. Le ministre d'État a obtenu une réduction de 30 % des importations d'huile de palme, et

Ma question s'adresse à M. Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics. Nous venons d'apprendre par la presse que Bercy, après la réunion d'un groupe de travail sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises, renonçait à réformer celle-ci. Si cette position se révélait exacte, elle serait grave, car elle voudrait dire que l'État n'a pas pris la mesure de l'injustice créée par l'évolution de la doctrine fiscale de l'administration. qu'il s'agit bien de cela : nous sommes nombreux à avoir été saisis soit par des vignerons pour des activités de pressurage à façon qui requalifient l'ensemble de leurs installations alors même qu'elles ne sont pas concernées par une activité de prestation, soit par des entreprises dont les entrepôts sont requalifiés au motif qu'il y a, par exemple, un chariot élévateur ou trop d'emplois sur le site. Monsieur le ministre, ces requalifications sont dues non pas à un changement de texte, mais à un changement de doctrine de l'administration fiscale, qui, d'ailleurs, comme pour s'en excuser, prétend que c'est à la demande des collectivités locales que cette évolution est faite, ce qui est faux- je ne connais personne qui aurait formulé cette demande. Monsieur le ministre, ma question est double : avez-vous vraiment renoncé à revenir sur ces évolutions doctrinales ? Si oui, comment justifiez-vous cette position contraire à une politique favorable à l'efficacité économique ? quelles avancées ont été effectuées, qui pourraient rassurer le monde viticole par ailleurs bien malmené dans les conditions climatiques actuelles et les entreprises qui ont vu parfois leur taux d'imposition multiplié par quatre

je vais essayer de vous rassurer sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises née après la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Conformément aux engagements pris lors des débats sur la loi de finances pour 2018, le Gouvernement clarifiera dès cet été la réglementation concernant la qualification industrielle ou commerciale des locaux professionnels. De plus, une première série de mesures législatives sera présentée au Parlement lors de la discussion de la prochaine loi de finances pour encadrer et préciser davantage le régime applicable et mieux accompagner les entreprises. Un groupe de travail a été mis en place début février pour élaborer ces propositions, et non pas, comme vous semblez le craindre, pour abandonner cette réforme. Ouvert aux représentants des entreprises et des associations nationales de collectivités territoriales, ce groupe de travail technique a permis de faire un état des lieux des difficultés rencontrées par certaines entreprises, notamment les entreprises artisanales, agricoles ou logistiques que vous avez citées, et ce à la suite de contrôles requalifiant leurs locaux professionnels en locaux industriels, entraînant ainsi des ressauts d'imposition en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises. Des propositions pour une réforme plus en profondeur de ce régime ont été formulées et doivent faire l'objet d'une évaluation plus complète et c'est pourquoi le groupe poursuivra ses travaux afin d'instruire ces propositions. L'ensemble de ces propositions sera présenté dans le rapport qui sera remis au Parlement d'ici au 1 juillet prochain. Par ailleurs, des instructions ont été données aux services fiscaux pour qu'ils fassent preuve d'un plus grand discernement dans le cadre de leurs contrôles en attendant que le nouveau cadre législatif soit défini. Aussi, je vous le confirme, nous irons bien au bout du travail sur l'évolution de la cotisation foncière des entreprises.

doute en aucun cas des qualités éminentes du préfet Morvan, mais je doute encore moins des qualités, de l'expérience et de la connaissance des problématiques territoriales de Philippe Bas, de Mathieu Darnaud et de Bruno Retailleau En écoutant les explications de notre collègue, un doute m'a pris : la mission première du Sénat n'est-elle pas de légiférer ? C'est une véritable question ! Les différents épisodes plutôt pathétiques, relativement récents, qui ont eu lieu dans cet hémicycle, sur lesquels je ne reviendrai guère, et dont on a parlé tout à l'heure- revalorisation des petites pensions agricoles, transfert des compétences eau et assainissement tout de même question ... Le Gouvernement et les « Marcheurs » n'aiment visiblement pas le débat parlementaire, sauf quand il vient de lui ... Absolument ! Mes chers collègues, un pays où l'on veut faire taire le Parlement, un pays où l'on veut faire taire tout court- on va bientôt examiner la loi sur les -est un pays qui a du souci à se faire. Je ne voterai pas cette motion, tout simplement parce que je préférerai toujours une république parlementaire à une « technocrature », fût-elle jupitérienne. M. Yves Détraigne, pour explication de vote.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

attachés profondément à cette république des territoires initiée par les lois de 1982, il nous appartient pleinement de prévenir toute forme de recentralisation et de favoriser la liberté locale et la cohésion territoriale. Or, si nous partageons l'idée qu'il est nécessaire d'apporter des correctifs aux dernières réformes territoriales, de la loi MAPTAM jusqu'à la loi NOTRe, nous partageons moins la méthode employée, qui a eu pour corollaire inéluctable de produire des réponses insuffisamment abouties.

respirer et s'organiser grâce à une intelligence territoriale qui a fait ses preuves. En définitive, nous devons faire confiance aux territoires. Toutefois, la méthode et la réelle finalité de ce texte posent question. question. Cette proposition de loi donne trop le sentiment d'avoir été déposée avec de la précipitation, heurtant ainsi la tempérance qui caractérise les travaux du Sénat.

tarde à arriver ? Pourquoi ne pas attendre la restitution, au début de juillet, des travaux du groupe de travail sur le statut des élus locaux, afin d'envisager un éventail complet et cohérent de mesures, qui protège les élus et qui réponde à la crise démocratique et à celles des vocations ?

Je l'ai indiqué précédemment, des ajustements utiles ont pu être trouvés, avec notamment les interventions du département en matière agricole, l'assouplissement des groupements de commandes pour les EPCI ou les mécanismes de fonds de concours, l'abaissement de la participation minimale des communes de moins de 1 000 habitants au financement des équipements publics, ou encore l'intérêt évident qu'il y a à renforcer le rôle de la région en matière d'emploi, de formation et de recherche, En revanche, cette proposition de loi revient sur des arrangements qui viennent d'être trouvés et qui se stabilisent. Elle induit des risques institutionnels, notamment par la généralisation de sortie à la carte des EPCI, et des risques fonctionnels, dans les arrangements qui viennent d'être trouvés entre les régions et les départements. En ce qui concerne les EPCI, on peut s'interroger sur la valeur des « pôles territoriaux », alors qu'un éventail d'outils considérables existe déjà et a été mis en place par les territoires. Si une nouvelle gouvernance doit s'imaginer au sein des EPCI, nous pensons qu'elle passe par davantage de liberté d'organisation du bloc local, avec la définition d'un principe de subsidiarité pour réguler les compétences. Toujours en ce qui concerne les EPCI, les conditions de retrait des communes membres constituent, sinon un risque de dépeçage, du moins un risque de déstabilisation et une remise en cause des politiques publiques mises en oeuvre. Je laisserai mon collègue Didier Marie compléter, et avant de conclure je citerai deux dispositions qui partaient d'une bonne intention mais dont on peine à mesurer l'applicabilité, en l'absence de prise en compte sérieuse des enjeux financiers

Pour conclure, je regrette de dire que, si des correctifs ont été apportés, cette proposition de loi, qui aura toujours le mérite de favoriser le débat, touche à des problèmes de fond mais s'apparente pour l'instant à un essai manqué.

de compléter à la marge la décentralisation et de proposer la création d'une agence pour la cohésion des territoires. Je commencerai par examiner cette dernière proposition. La création d'une agence pour la cohésion des territoires est une proposition sénatoriale, cela a été dit. Le Président de la République a d'ailleurs manifesté son intérêt pour cette formule lors de la Conférence nationale des territoires, l'année dernière. J'y vois plusieurs intérêts. Premièrement, agence permettrait de fédérer les acteurs de l'administration déconcentrée et des collectivités pour répondre aux besoins des territoires dans le domaine des soins, de l'accès aux services publics, de la mobilité et de l'accès au numérique. Deuxièmement, comme l'a rappelé voilà quelques semaines le commissaire général à l'égalité des territoires, elle pourrait venir appuyer les territoires en difficulté en matière d'ingénierie territoriale. Enfin, troisièmement, elle devrait devenir un véritable guichet unique pour les élus dans un souci de simplification des procédures et des conseils. Néanmoins, mes chers collègues, plusieurs questions se posent : quelle articulation avec le Commissariat général à l'égalité territoriale ? Quelle complémentarité avec la banque des territoires de la Caisse des dépôts et consignations, inaugurée il y a quelques jours ? En outre, je rappelle que notre assemblée est sur le point de créer une agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs, dans le cadre de la proposition de loi de nos collègues Rémy Pointereau et Martial Ne créerions-nous pas alors un doublon ? Enfin- cette question s'adresse à Mme la ministre -, quand pourrons-nous avoir accès au rapport de Serge Morvan sur la mise en place d'une telle agence ? Je rappelle que ce rapport était attendu le 15 mai dernier Pour conclure sur ce point, je crois que nous avons là une bonne idée, mais qui demanderait à être affinée, mieux articulée avec les dispositifs existants et qui ne doit surtout pas se transformer en une nouvelle usine à gaz- je ne doute pas que notre assemblée saura faire preuve de vigilance sur ce point. les autres dispositions de cette proposition de loi, j'estime que la volonté d'aménager et de corriger la réforme issue de la loi NOTRe est une bonne chose. En matière de réforme territoriale, il nous faut maintenant ajuster, et non plus brusquer. En effet, les élus locaux ont assez des grands soirs territoriaux qui amènent toujours leur lot de complications. Comme notre commission des lois le dit souvent, laissons respirer nos territoires. Cela dit, la respiration n'exclut pas des ajustements, ceux qui sont relatifs aux compétences des départements. Ils vont dans le bon sens ; le renforcement de la capacité d'intervention des départements en faveur de l'agriculture et de la pêche et leur contribution au financement des opérations d'investissement permettront d'étoffer leur compétence de solidarité et de cohésion territoriale. les dispositions consacrées aux coopérations intercommunales, la plupart des éléments vont dans le sens d'une plus grande liberté et c'est heureux. En ce qui concerne l'échelon régional, je partage le constat des auteurs c'est une aberration de maintenir une cloison étanche entre, d'un côté, les politiques d'apprentissage et de formation professionnelle, qui relèvent en grande partie des conseils régionaux et, de l'autre, la politique de l'emploi, qui demeure centralisée. crois que les régions ont déjà des outils pour faire des choses utiles. Prenons l'exemple de ma région, les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, son président, a mis en place des dispositifs extrêmement innovants, qui sont complémentaires complémentaires de Pôle emploi et de l'action de l'État, en créant la plateforme Proch'emploi, qui a permis à 10 000 personnes de trouver un emploi, en mettant en place un « Pass Formation des aides aux transports, ou encore en signant un partenariat avec Linkedln pour développer des outils numériques. Et ce ne sont là que quelques exemples. Alors, oui, on peut donner à la région un rôle de coordination des services et lui déléguer davantage de compétences, mais, vous le voyez, on peut faire beaucoup plus avec ce qui existe déjà. Enfin, nous soutenons totalement les dispositions qui visent à améliorer la condition des élus et à rendre plus attractif l'exercice des mandats locaux. En la matière, il faut marcher sur deux jambes : à la fois simplification des sujétions et des formalités, et hausse des gratifications. Nous espérons que le Gouvernement entendra ces deux nécessités pour rendre au mandat d'élu local ses lettres de noblesse. Cette proposition de loi est donc équilibrée et mesurée. On constate qu'elle recoupe plusieurs initiatives en cours. J'espère que nous parviendrons à fédérer toutes les énergies pour améliorer la cohésion de nos territoires et l'exercice de notre démocratie. J'appelle le Gouvernement, madame la ministre, à prendre en compte les propositions du Sénat, qui est ici dans son rôle le plus légitime et le plus sacré, celui de la défense des territoires et des collectivités.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est à l'aune de la vitalité de la démocratie locale que l'on mesure l'état démocratique d'une nation. Tocqueville faisait ce constat dès 1830 en écrivant que c'est « dans la commune que réside la force des peuples libres » et en ajoutant que « sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté Les promoteurs de la loi NOTRe ont-ils lu Tocqueville ? Permettez-moi d'en douter, tant l'édifice territorial tel qu'il résulte des lois adoptées ces dernières années ne paraît pas contribuer à vitaliser la démocratie de proximité, en raison de l'éloignement toujours plus grand des instances de décision et de l'émergence d'une technocratie locale. sommes ou que nous avons été le savent, la mise en oeuvre de ces lois ne s'est pas faite sans heurts. Le Parlement a d'ailleurs adopté plusieurs aménagements nécessaires, venant ainsi assouplir les rigidités initiales. Je pense notamment à la proposition relative à l'élection des conseillers métropolitains, adoptée sur l'initiative du groupe du RDSE et portée par notre collègue Mireille Jouve. Si l'on fait l'état des lieux de l'intercommunalité telle qu'elle est aujourd'hui, on constate que les élus ne s'y retrouvent pas. Le découpage territorial et la nouvelle répartition des compétences, s'ils pouvaient relever d'une certaine logique, résistent mal à l'expérience concrète, à la réalité de nos territoires. Par exemple, l'intercommunalité de 16 000 habitants où je siège toujours doit aujourd'hui, du fait des transferts de compétences qui relevaient autrefois du département, cautionner des emprunts sur les stations de ski pour des montants exorbitants. On fait donc face à des élus désarçonnés, pour ne pas dire désabusés, devant des transferts qui les dépassent parfois. On se retrouve aussi avec des intercommunalités qui, pour maintenir un équilibre avec les plus petites communes qui les composent, ne peuvent pas ou ne peuvent plus se consacrer à l'objet qui fut le leur à leur création, le développement économique de leur territoire. Le présent texte vise à apporter des ajustements, vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur- je tiens d'ailleurs à souligner votre travail, précis et pragmatique. Je note toutefois que certains de ces ajustements sont d'ampleur. Aussi, plusieurs dispositions de la proposition de loi suscitent notre approbation. Par exemple, l'article 9 ouvre la porte à un exercice territorialisé des compétences intercommunales dans des EPCI de taille « XXL ». Il répond à une logique de subsidiarité et à une demande exprimée sur nos territoires. En ce qui concerne le département, si la question de son maintien s'est posée en son temps, il reste et demeurera un échelon essentiel de proximité, de solidarité et d'action dans nos territoires. Ainsi nombre de mes collègues du RDSE et moi-même nous retrouvons-nous dans les articles 12 à 15, de manière très concrète, que ce soit en matière d'aménagement ou de soutien aux activités agricoles. Ces dispositions permettent à nos départements d'être pleinement reconnus dans leur rôle de solidarité territoriale. Partisans d'une véritable décentralisation, nous sommes aussi favorables à un renforcement des compétences des régions en matière d'emploi, trop peu développées aujourd'hui, ou en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Néanmoins, si nous pouvons souscrire à certaines dispositions prévues dans ce texte, cette proposition nous met mal à l'aise. J'entends ce que nous disent les élus, ils ont dû mettre en oeuvre les récentes lois de réforme territoriale, les digérer ; ce ne fut pas toujours simple. Ils nous réclament donc aujourd'hui de la stabilité et nous demandent de ne pas modifier sans cesse la législation. Or comment ne pas voir, par exemple, dans l'article 10 une source d'instabilité ? prévoit un mécanisme permettant à plusieurs communes d'un EPCI, sous réserve de remplir plusieurs critères, de « faire sécession » dudit EPCI et d'en créer un nouveau. On déferait donc des EPCI qui viennent d'être achevés, parfois non sans mal ? On remettrait en cause des compétences qui ont déjà été transférées Le risque d'incompréhension des élus, mais aussi de nos concitoyens, est grand. De plus, nous considérons cette proposition comme un texte d'appel, réalisé de manière précipitée, ce qui n'est pas l'habitude de la Haute Assemblée.

Nous pouvons tirer les mêmes conclusions concernant les articles du titre I créant une agence nationale pour la cohésion des territoires. Sur toutes les travées, nous le savons, la création de cette agence, annoncée voilà près d'un an par le Président de la République, ici même, au Sénat, est en cours. Ses contours, ses champs d'action, ses financements et son insertion dans le paysage institutionnel doivent encore faire l'objet d'arbitrages. La question des communes nouvelles était également inscrite dans le texte initial. L'article 8 visait à prolonger, déraisonnablement à notre sens, les dérogations en matière de représentation des communes déléguées au sein d'EPCI. Nous le savons, notre collègue Françoise Gatel, dont l'expertise en la matière n'est plus à prouver, prépare un texte plus général visant à améliorer la législation applicable aux communes nouvelles. C'est pourquoi nous avons soutenu la suppression de cet article 8. ce texte réunit un ensemble disparate de dispositions, dont certaines pourraient recueillir notre approbation. Nos territoires mériteraient aujourd'hui que l'on analyse en profondeur et sans précipitation, à l'occasion d'un important travail de fond, leurs difficultés à mettre en place de vrais outils de développement et de service pour nos concitoyens.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, sur toutes les travées, nous convenons régulièrement que nos territoires ont d'abord besoin de visibilité, donc de stabilité, bref, qu'on leur fiche la paix. Oui ! Les sujets abordés de manière partielle au travers de cette proposition de loi, en matière de formation, d'apprentissage, d'emploi, de responsabilité et de statut des élus, de simplification de la vie et de l'organisation des territoires, mériteraient chacun un texte ou une démarche approfondie, globale, donnant durablement la visibilité tant attendue. Or des travaux de fond sont engagés sur tous ces sujets par ailleurs. Pas sur le département ni sur la région ! Il ne s'agit donc pas de répondre au calendrier du Gouvernement, mais simplement de bénéficier des travaux et de discuter sur le fondement de propositions, et non seulement sur le fondement de celles qui sont attendues. De ce point de vue, l'opportunité de ce texte nous semble discutable. Nous ne souhaitons pas compromettre ces travaux de longue haleine, initiés notamment au Sénat.

La suppression de l'obligation de réalisation d'un schéma et de ses orientations n'est pourtant pas souhaitable. Par ailleurs, ce texte supprime l'obligation de déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. Pourtant, l'obligation de déclaration de candidature est une garantie de la lisibilité et de la sincérité du scrutin. Elle harmonise la règle de droit avec les autres élections sans pour autant porter atteinte à la liberté de candidature, ... C'est mal connaître les communes rurales ! ... car il est possible dans les communes de moins de 1 000 habitants de faire des candidatures groupées Surtout- nous sommes tous sensibles à cet argument, qui a fait l'objet de nos débats et d'un vote unanime récemment -, elle permet d'éviter les « candidats malgré eux N'était-ce pas le sens de notre démarche lorsque nous avons adopté, en janvier dernier, la loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections ? L'article 17 confie à la région le soin de coordonner les acteurs des politiques de l'emploi, pour une territorialisation accrue de ces politiques, et de consolider les compétences régionales

Pourquoi se priver d'une approche plus complète et plus au service de nos territoires et de notre action publique ?

Ainsi, comme j'ai pu le dire en commission, alléché par le titre de la présente proposition de loi, j'aurais souhaité un traitement de la loi NOTRe autre que les soins palliatifs qui nous sont proposés. sont utiles, en ce qu'ils rendent plus supportables les effets de ladite loi sur les collectivités et leurs élus, mais ils ne font que retarder l'heure où l'on réalisera pleinement ce que cette loi a de mortifère et où l'on prendra conscience qu'il faut purement et simplement la supprimer. On me dit que les élus sont las de l'instabilité du code général des collectivités territoriales et qu'ils rêvent d'une pause qui leur permettra de reprendre leur souffle.

-de rêver de n'être plus obligés de faire de manière compliquée, au moyen de bricolages locaux, ce qu'ils feraient simplement et généralement volontiers, sans la camisole de force qu'on leur a imposée.

priver les communes de leur liberté de s'associer, de décider de la taille de leurs intercommunalités et d'en négocier les statuts, le tout sur fond de contraintes budgétaires et d'odes au gigantisme, censé apporter la solution aux difficultés aux difficultés artificiellement créées. Priver les départements de la liberté d'aider qui ils veulent et selon les modalités qui leur semblent les plus adaptées à leur territoire et à leurs moyens, voilà la tendance lourde, qui, du cela, je serais mal venu de nier que cette proposition de loi desserre un peu la camisole imposée aux élus. Ne reste plus qu'à espérer que nos débats permettront d'aller un peu plus loin, s'agissant notamment de l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux, particulièrement des mandats municipaux dans les plus petites collectivités. Admettez, mes chers collègues, que la proposition de loi passe un peu vite sur cette question, particulièrement importante et sensible ! Combien de fois n'en avons-nous pourtant pas discuté ici ? ici ? L'essentiel des autres dispositions, dont beaucoup ont, d'ailleurs, déjà été adoptées par le Sénat, faciliteront certainement la respiration des territoires. Par exemple, l'article 9 officialise la création de « pôles territoriaux traitement léger des troubles du gigantisme. L'article 10 donne la possibilité à des communes, sous certaines conditions, de migrer vers un autre EPCI. EPCI. Les articles 12, 13, 14 et 15 donnent plus de libertés aux départements pour exercer la solidarité territoriale. L'article 22 légalise la subdélégation de la compétence transports scolaires transférée par la région.

Quant à l'article 8, relatif aux communes nouvelles, notre commission a bien fait, selon moi, de le supprimer. Autant la création d'une commune nouvelle entre des collectivités proches, partageant les mêmes préoccupations et pratiquant déjà souvent la mutualisation des moyens, est de simple bon sens, autant la fusion de communes souvent disparates motivée par les seuls avantages financiers qu'on leur a fait miroiter, créera plus de problèmes qu'elle n'en réglera. Tout à fait ! En tout cas, je ne vois pas pourquoi ces communes continueraient à bénéficier de dotations majorées ou maintenues au détriment des autres en même temps qu'elles conserveraient la représentation plus avantageuse des communes anciennes au conseil communautaire. Un peu de logique ! Si l'on crée une commune nouvelle, c'est avec les avantages et les inconvénients du statut des communes nouvelles.

qui nous ont été imposés et dont je ne comprends toujours pas l'utilité. Incontestablement, la fabrication de « schémas » occupe les bureaux et les élus ... Pour le reste, ils ont surtout la capacité d'empêcher de faire. Quant à « l'Agence nationale pour la cohésion des territoires », elle vient opportunément masquer le désengagement de l'État des territoires. Certes, une agence, c'est mieux que rien, mais cela ne remplace pas une politique de cohésion territoriale de long terme, dotée de moyens financiers et humains à la hauteur des enjeux. Il est fâcheux que la France se mette à généraliser ces modèles de gestion territoriale au moment où leurs promoteurs initiaux en Europe, les Britanniques, commencent à en voir les limites et les effets politiques calamiteux.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : polissez-le sans cesse et le repolissez ; ajoutez quelquefois, et souvent effacez », cette célèbre maxime de Boileau trouve ici toute son illustration. Nos collectivités ont connu, au cours des dernières années, de très nombreuses réformes, de trop nombreuses réformes. Je me permets de vous rappeler, mes chers collègues, qu'un rapport d'information très récent de notre assemblée, mars 2017, portait le titre. Nos collègues du groupe Les Républicains nous proposent aujourd'hui d'« apporter des correctifs indispensables » aux dernières réformes territoriales, qui sont « d'inspiration technocratique, adoptées précipitamment et appliquées parfois avec brutalité ».

au-delà du constat, cette proposition nous invite à rebattre les cartes, même si les auteurs nous assurent qu'« il n'est évidemment pas question [ ...] de bouleverser à nouveau l'architecture institutionnelle de nos territoires En effet, des modifications assez substantielles sont proposées pour quasiment chaque niveau de collectivités. Communes, intercommunalités, départements et régions, tout le monde a droit à ses aménagements. Je ne vais pas, à ce stade, revenir sur chacune des mesures proposées, M. le rapporteur l'ayant brillamment fait précédemment. Globalement, bien sûr, certaines d'entre elles paraissent séduisantes, mais nous n'oublions pas l'écueil que nous tentons régulièrement d'éviter : trop de lois, trop de changements, sans même avoir eu le temps d'en évaluer la pertinence avec un minimum de recul. Là est sans doute la question.

Je peux en témoigner, puisque c'est précisément le cas sur mon territoire, avec la communauté urbaine du Grand Reims, qui rassemble 206 élus, représentant 143 communes, sans que nous ayons ressenti le besoin de nouvelles modifications législatives. L'expérience fonctionne, et personne ne demande à en sortir.

de notre rapporteur, qui nous explique que ce schéma n'est pas prescriptif et qu'il a fait son temps. Mais je vois aussi que le schéma de coopération intercommunale est très symbolique. On peut d'autant plus s'interroger sur sa suppression,

Je veux ensuite évoquer le titre I du texte. Celui-ci crée une agence nationale pour la cohésion des territoires. Sans m'appesantir, sur le fond, sur le rôle de la nouvelle agence, je souhaite tout de même faire une remarque de forme. Sauf erreur de ma part, le Sénat s'apprête à voter, au cours de la même semaine, au sein de propositions de loi différentes, la création de deux agences nationales. En effet, notre Haute Assemblée de la proposition de loi de nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin, qui prévoit notamment la création d'une agence nationale pour les centres-villes et centres-bourgs.

a peu, est-ce bien indispensable, surtout après le texte que j'évoquais à l'instant ? Sur le fond, j'ai encore un peu plus de mal à comprendre, puisque le texte de la commission prévoit expressément que l'Agence nationale pour la cohésion des territoires sera compétente pour la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes.

et n'ayons pas peur des initiatives venant du terrain, y compris en matière d'intercommunalité. Comme plusieurs de mes collègues du groupe Union Centriste, je serai attentif à l'évolution du texte en séance publique. La parole

Le mandat municipal 2014-2020 est compliqué et difficile pour nombre d'élus, qui, lorsqu'ils ont accédé aux fonctions de maire, adjoint ou conseiller, n'imaginaient pas devoir faire face à de tels changements. Bien évidemment, le bouleversement territorial effectué ces dernières années est très loin d'être parfait et a souvent été conduit avec une forme de brutalité et beaucoup d'incohérence. La carte des régions, dessinée sur un coin de table, est totalement hétérogène, avec de très grandes régions et d'autres restées dans leur plus petit périmètre. La suppression du conseiller territorial, qui créait un lien singulier mais efficace entre région et département, a été une grossière erreur, fruit d'une inutile arrogance. Quant à la multiplication de métropoles, je suis extrêmement dubitative car elles ne correspondent pas à la réalité d'une vraie métropole. On pourrait citer bien d'autres exemples. Comme mes collègues du Maine-et-Loire, je représente un département « hors normes » par l'ampleur de la recomposition territoriale depuis 2013, date de naissance de la première commune nouvelle, celle de Baugé-en-Anjou. En 2012, le département comptait 363 communes. Au 1 janvier 2018, il n'en dénombre plus que 184, soit une réduction de 47,6 %. communes sont envisagées. La carte des EPCI s'est elle aussi modifiée, passant de trente à neuf intercommunalités, dont une communauté urbaine et trois communautés d'agglomération. Je sais que beaucoup s'effraient ou, du moins, s'interrogent sur une telle évolution. Mais il faut rappeler que celle-ci est le fruit d'une histoire de coopération ancienne entre les communes. La dernière et seule commune à être entrée en intercommunalité l'a fait il y a plus de vingt ans. Les élus ont des habitudes de travail en commun, qui se traduisent par des communautés de communes pour certaines très intégrées. L'exemple le plus abouti est celui des Mauges, où six communautés de communes, au sein d'un pays dynamique, sont devenues six communes nouvelles

Mais il est vrai que cela n'est pas un long fleuve tranquille, et loin de moi l'idée de reprocher aux communes qui avancent à leur rythme ou qui souhaitent demeurer communes historiques de ne pas accélérer. Ce que je veux affirmer, c'est qu'il faut aussi répondre à ceux qui sont allés loin dans la recomposition sur la base d'un projet territorial fort, et pas seulement attirés par l'appât financier de dotations préservées. Nos EPCI, en Maine-et-Loire, dépassent très largement le seuil démographique imposé par la loi. Certaines intercommunalités n'ont pas souhaité rester à ce seuil et ont fusionné, ce qui a aussi encouragé la création des communes nouvelles.

Dans le texte de ce jour, je me réjouis que la commission des lois ait supprimé l'article 8, qui prolongeait la dérogation relative à la représentation des anciennes communes d'une commune nouvelle au sein d'un EPCI. Autant une période transitoire était nécessaire, autant une prolongation serait un mauvais signal et un facteur de déséquilibre. Vous m'avez rassurée, monsieur le rapporteur, quant à l'article 10, qui nous inquiétait, mon collègue Stéphane Piednoir et moi, sur le risque d'instabilité qu'une scission au sein d'un EPCI nouvellement créé pouvait faire naître. Je sais Je sais que, dans nombre de départements, sous la pression des représentants de l'État, des mariages forcés et imposés aux élus créent des difficultés majeures. Vous avez confirmé que des garanties entouraient l'article 10. Nous vous faisons confiance sur ce point.

Concernant les articles relatifs au département et à la région, je tiens à faire deux remarques. Le problème actuel des départements est essentiellement lié à l'étranglement financier qui résulte des dépenses sociales décidées par l'État, mais financées par ce niveau de collectivités.

Cela ne vaut cependant pas quitus sur le texte, qui, sur le fond, nous laisse pour le moins perplexes. Concernant la méthode, alors que la majorité dénonce régulièrement et à juste titre l'usage intempestif de la procédure accélérée

étonnant que, dans le même temps, de multiples travaux sont menés par le Sénat pour évaluer l'impact des récentes réformes territoriales, revitaliser le rôle des communes, ajuster le fonctionnement des communes nouvelles, créer un véritable statut de l'élu ou encore redynamiser les centres-bourgs.

Dans le texte initial, vous en remettiez en cause des pans entiers, revenant notamment sur la relation entre commune et intercommunalité, en tentant de rétablir subrepticement la clause de compétence générale des départements ou en revenant sur le chef de filat de la région en matière économique ou de transport. Vous prenez là le risque de déstabiliser un édifice qui est en cours de consolidation et qui a besoin d'une pause et d'une respiration. Ce texte, à nos yeux prématuré et précipité, a tout de même été remanié et, pour partie, vidé de ses dispositions les plus discutables Nous pouvons ainsi saluer la sagesse de M. le rapporteur, qui a proposé la suppression de l'article 8, lequel surreprésentait jusqu'en 2032 les communes nouvelles dans les EPCI,

vous avez maintenu le titre I, créant une agence nationale pour la cohésion des territoires. Cette agence est attendue. Nous en soutenons le principe pour remédier aux fractures territoriales, mais, là encore, la précipitation n'est pas bonne conseillère et nous savons toutes et tous que le nouveau

Il en est ainsi de ceux qui facilitent le retrait de communes d'un EPCI, de la nécessaire déclaration de candidature de tous les prétendants au suffrage universel des communes de moins de 1 000 habitants, de l'alourdissement des ordres du jour des conseils municipaux, des conditions de mise en oeuvre des délégations de compétence, de l'élargissement du droit de timbre sur les permis de construire et d'autres, sur lesquels nous reviendrons pour exprimer notre désaccord. Ce texte touche-à-tout, composé de dispositions diverses, pas nécessairement inutiles pour certaines, mais très loin de l'ambition simplificatrice affichée par les signataires, risquerait, s'il était adopté, de produire l'effet inverse de celui qui était recherché et, plutôt que de répondre aux interrogations et inquiétudes de certains élus, ne ferait qu'accentuer leurs difficultés, par une législation à la hâte. Nous avons besoin de stabiliser l'édifice territorial, révolutionné par les lois MAPTAM et NOTRe. Nous avons besoin de faire une pause, d'évaluer la nouvelle architecture et d'en corriger, le moment venu, les imperfections.

madame la ministre, mes chers collègues, l'équilibre territorial sera évidemment un enjeu crucial pour notre pays dans les années et les décennies à venir. je ne peux personnellement que soutenir cette proposition de loi, visant à remédier à la fracture grandissante entre des territoires urbains et les secteurs périphériques, banlieues, bourgs et campagnes, qui sont les laissés-pour-compte de la métropolisation. Madame la ministre, vous le savez, il n'y a plus depuis longtemps en France de politique d'aménagement du territoire et, bien que je me méfie de la

cette agence ne servira à rien si elle reste une coquille vide, ce qui m'oblige à répéter ce que nous, les Républicains, avions défendu lors de la dernière campagne législative, que, pour un euro investi dans les banlieues, un euro doit être investi dans la France des petites villes et des villages, qui est en train de mourir lentement mais sûrement. ! Le pire, dans l'affaire, est que le processus d'intercommunalité, souvent présenté comme étant le gage de survie de ces territoires, est en train d'assécher ces derniers et de les priver de leur substance, au profit des centres-villes. Je dénonçais déjà ce phénomène déjà ce phénomène voilà douze ans, dans Si l'on veut sauver nos territoires, si l'on veut trouver encore des élus locaux, demain, pour gérer nos communes rurales ou celles de banlieue, il faut aller dans le sens de cette proposition de loi. Il faut restaurer la confiance, il faut redonner des marges de manoeuvre aux maires, leur permettre de choisir au lieu de subir, réinstaurer le droit à l'expérimentation afin de fédérer les énergies et faire émerger les projets d'avenir, car ce sont les élus locaux, qui, au quotidien, sont les aménageurs du territoire. Finalement, qu'est-ce qui prouve qu'une grande taille est une assurance d'efficacité ? C'est peut-être vrai dans le monde des affaires, mais l'histoire a toujours démontré que les plus grands empires étaient les plus fragiles ! D'ailleurs, dans le domaine hospitalier, on nous demande aujourd'hui de recréer de petites unités pour sauver les urgences. Craignons que cet affaiblissement ne se produise aussi pour nos collectivités. À propos de l'Île-de-France, nos gouvernants n'ont qu'un mot à la bouche, dont ils se gargarisent, la « métropole », avec, autour d'elle, une idée reçue : un territoire concentrant toutes les richesses et tous les potentiels. Or, derrière les mots, la réalité est souvent bien bien différente : la banlieue n'est pas Paris, la Seine-Saint-Denis est presque aussi riche que les Hauts-de-Seine et la moitié de la surface de l'Île-de-France est consacrée à l'agriculture. On est loin de l'image que l'on donne Avec les lois NOTRe et MAPTAM, nous subissons un désordre territorial kafkaïen qui étouffe les communes, bride les initiatives et enferme les élus locaux dans une toile d'araignée qui les paralyse de façon insidieuse.

donc du développement économique de nos communes. À ce rythme, nous n'aurons bientôt plus que les chrysanthèmes à inaugurer ... Pour conclure, je Pour conclure, je suis heureux de soutenir cette initiative, qui vise à restituer un cadre à l'aménagement du territoire, à donner, je l'espère, plus de souplesse aux élus locaux et à corriger certains déséquilibres institutionnels, nés de la prolifération de réformes de l'organisation territoriale de ces dernières années. J'irai même plus loin : au moment où il faudrait que nous attendions, le petit doigt sur la couture du pantalon, que M. le Président de la République daigne nous confier quelle organisation territoriale aurait ses faveurs, alors même- et c'est peut-être notre drame -qu'il n'a jamais été un élu de proximité, ne serait-il tout simplement pas de bon sens de revenir à une organisation à trois strates, avec une région métropole,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet de l'équilibre territorial et de la vitalité de la démocratie locale est primordial.

Cette nouvelle forme est non seulement dangereuse pour l'équilibre territorial- il suffit de regarder les différences de soutien de l'État pour les villes et pour les campagnes -, mais emporte aussi une conséquence désastreuse pour l'avenir : un manque de pragmatisme et de bon sens qui conduit le Gouvernement à prendre des décisions fâcheuses pour l'avenir de nos territoires. Dernièrement, la problématique du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités en a été un malheureux exemple : malgré les alertes répétées des élus ruraux, rien n'a changé. L'obstination jacobine et technocratique a sévi. Seuls quelques aménagements à la marge ont été concédés pour faire avaler la pilule, mais le fond est resté le même : dépouiller les communes des compétences qu'elles ont toujours exercées afin de les affaiblir refuser de les laisser choisir à partir de leur connaissance du terrain. Il serait pourtant si simple de faire plus confiance aux élus locaux, de les laisser gérer leur destinée. N'oublions jamais qu'à la suite de la Révolution française, c'est le peuple qui a voulu que la commune soit créée et qu'elle soit administrée par des élus issus de ses rangs. D'ailleurs, ne nous y trompons pas : de tous les élus, le maire est le plus plébiscité par les Français, dans tous les sondages. Car nos maires sont la proximité. Cette proximité dont a besoin tout un chacun pour se sentir écouté et entendu. Cette attente de proximité, c'est aussi la bonne gestion de l'argent public en dépit de contraintes budgétaires toujours plus fortes. C'est encore et surtout la capacité de nos maires à gérer l'intérêt général, sans jamais oublier que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers.

Il faut absolument redonner du courage à nos élus en les respectant, en les associant et en leur faisant confiance. Pour nos territoires ruraux, chaque échelon territorial a son importance. Aux côtés des communes, les départements sont aussi des acteurs de l'équilibre territorial. Dans notre Dans notre pays, traversé par des fractures, ils sont aussi un réel échelon de proximité. Leur rôle s'est amplifié sur les missions de solidarité humaine. Aussi, il me paraît essentiel de rationaliser l'ensemble de l'action sociale familiale sur cet échelon, en fusionnant les caisses d'allocations familiales avec les départements. Cette mesure permettrait une gestion coordonnée de cette politique publique à un niveau pertinent et une meilleure gestion de l'argent public. L'aménagement des territoires fait aussi partie des missions départementales. Il serait ainsi légitime, comme je le propose dans un amendement, de transférer, avec les moyens afférents, l'entretien des routes nationales aux départements qui le souhaitent, pour les tronçons qui les traversent. Pour conclure, Pour conclure, madame la ministre, je dirai que la France des 36 000 communes n'est pas ringarde. Absolument ! Nous n'avons pas besoin de copier d'autres modèles : le nôtre est le fruit de notre histoire, le fruit de femmes et d'hommes qui ont lutté pour notre idéal de liberté, d'égalité, de fraternité. Ne l'oublions pas. N'oublions pas non plus les fantassins de la République que sont les élus locaux. Ce

la future agence nationale pour la cohésion des territoires aurait pour rôle principal d'être l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales en matière d'ingénierie humaine et financière pour l'ensemble des projets, des investissements et des expérimentations.

Néanmoins, les fusions envisagées ne doivent pas amoindrir les ressources de ces structures déjà mises à mal dans la précédente loi de finances. Il faut être cohérent. Si l'on veut accompagner correctement les projets des collectivités, il faudra des moyens humains et financiers. De l'égalité à la cohésion des territoires, que dissimule ce glissement sémantique ? Quelle complémentarité existe-t-il avec l'action des départements ? La banque des territoires a été mise en place le 30 mai dernier. Elle est déjà opérationnelle dans deux départements. Quelle sera son articulation avec la nouvelle agence ou encore avec La Poste ? Nous attendons aussi le rapport de M. Serge Morvan, nouveau commissaire général à l'égalité des territoires, qui devrait être remis au Premier ministre pour la mi-juin. À ce stade, nous n'avons donc que très peu d'éléments. Le Gouvernement semble entretenir volontairement le flou sur les missions de l'agence. nous partageons l'impatience de nos collègues de la majorité sénatoriale sur le rôle de l'ANCT. Cette proposition de loi, malgré tous ses défauts d'écriture, permettra peut-être d'avoir quelques lignes directrices de l'action gouvernementale en direction des collectivités, mais j'en doute.

chambre des territoires, être méthodiquement écarté de toute concertation. Je pense que les sénateurs de tous bords auraient pu apporter une expertise judicieuse dans le domaine du développement territorial.

cohésion des territoires. Si elle va dans le sens d'une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs publics dans les territoires, objectif auquel votre rapporteur pour avis souscrit naturellement,

développement durable ? Cet amendement rédactionnel vise à insister sur la nécessité d'instaurer une stricte parité entre les hommes et les femmes dans la composition du conseil d'administration de l'Agence. La rédaction actuelle de l'article, telle qu'elle résulte des travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, satisfait cet objectif. En outre, elle reprend la formulation votée par le Sénat lors de la création de l'Agence française pour la biodiversité.

8 rectifié vise à rendre possible la suppression d'une partie seulement des communes déléguées. Aujourd'hui, dans la loi, soit on maintient toutes les communes

une partie seulement des communes nouvelles, sous réserve évidemment de l'accord des communes déléguées concernées qui pourrait se manifester soit par un vote du conseil municipal de la commune déléguée, lorsqu'il en existe un, soit, lorsque tel n'est pas le cas, par une consultation Cela apporterait une souplesse. J'ajoute que cela sécuriserait les communes déléguées, parce que, avec le système actuel, on a pu observer- je l'ai vécu notamment dans mon département -la possibilité pour un conseil de commune nouvelle

tout en maintenant les communes déléguées, de faire en sorte qu'il n'y ait pas systématiquement une mairie annexe dans chaque commune déléguée. Là aussi, c'est une demande qui émane du terrain. En effet, le maintien de mairies annexe a un coût-

Quel est l'avis de la commission ?

Trois ans et demi au cours desquels nous avons recueilli l'avis des maires, notamment sur le sujet des grandes intercommunalités, qui nous demandent

pour organiser des pôles de proximité. Nelly Tocqueville et moi-même sommes à l'origine de la création d'une grande intercommunalité, aujourd'hui métropole Rouen-Normandie. Dès l'origine,

qui est consultée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les modalités d'exercice des compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-3, et leur modification ainsi que sur tout sujet d'intérêt du pôle. » Je ne sais pas si vous percevez le caractère contraignant que tout cela induit ? Dans toutes les intercommunalités, en plus des commissions permanentes et des bureaux, il va y avoir des commissions va y avoir des commissions et des conseils de pôles. Dans un grand nombre de cas, on ne pourra prendre de décision pour les modalités d'exercice des compétences et pour tout sujet susceptible d'intéresser le pôle qu'après consultation de ce dernier. Je le répète : tout cela est extrêmement contraignant, et je préfère, comme l'a excellemment dit M. Kerrouche, la grande liberté qui existe aujourd'hui. Dans quantité d'intercommunalités, on a bien vu qu'il fallait s'organiser par secteur- c'est du bon sens -, mais faisons-le librement et simplement. La parole est

des lois. Sur notre territoire, qui est vaste, les situations peuvent être très différentes. Certains sont satisfaits de la manière dont fonctionnent les intercommunalités qu'ils ont volontairement constituées, que d'autres sont très insatisfaits d'intercommunalités que les préfets leur ont imposées. Nous voulons que ceux qui sont satisfaits le restent et que ceux qui sont insatisfaits le soient un peu moins. Il ne s'agit pas de forcer la main à qui que ce soit ! Toutefois, il n'est pas exact de dire que les pôles territoriaux figurent dans la loi. Quand ils existent, ce sont des arrangements. Si ces derniers donnent satisfaction, n'y touchez surtout pas, mais n'empêchez pas vos voisins

Les dirigeants de ces intercommunalités se trouvent contraints par l'excès de compétences qu'ils exercent. Pour autant, ils ne peuvent pas s'en affranchir, soit parce que les communes rurales ne peuvent pas les exercer, soit parce qu'il n'y a pas assez de communes nouvelles.

proximité de toute responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Nous voulons, avec beaucoup de modestie, fournir un outil supplémentaire, sans rien retirer à qui que ce soit.

75 % des élus du Pays basque ont voulu cette intercommunalité, devenue la communauté d'agglomération du Pays basque, et 75 % des conseils municipaux ont également opté pour cette intercommunalité XXL.

et demi. Je souhaite voir aboutir le travail que Mathieu Darnaud conduit, au nom de la commission des lois, sur l'évaluation

est maladroit et aura des conséquences perverses allant à l'encontre de ce qui est recherché, notamment dans le cadre d'une stabilité politique institutionnelle et territoriale.

explication de vote. Cet article pose un problème majeur. Il intervient à une période où l'édifice intercommunal est en train de se stabiliser.

Ce faisant, c'est l'ensemble d'un édifice qui sera fragilisé, mis à mal, alors que, face à de réelles difficultés, cela a été rappelé par plusieurs d'entre nous, il existe des procédures de droit commun permettant de sortir calmement

après un vrai débat démocratique, comme cela aurait dû se passer partout, se sont inscrits dans une volonté de regroupement. Ma crainte est forte - c'est la raison pour laquelle j'ai émis des réserves sur cet article et que je ne le voterai pas que, sur une petite partie d'un territoire d'une grande intercommunalité mise en place par la volonté des élus, ne se manifeste une intention de fragmentation en appelant d'autres. Je regrette que cet amendement de suppression et cet article ne prennent pas suffisamment en compte la différence entre les intercommunalités créées par la volonté des élus

la CDCI n'est consultée que pour avis dans cette procédure dérogatoire. Sans doute aurait-il été plus pertinent- j'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens

avons donc voté en responsabilité- croyez-moi ! -, en obtenant du gouvernement de l'époque un certain nombre d'améliorations. C'est le rôle du Sénat : ne pas être la chambre du refus, mais être au contraire une chambre qui protège les territoires

que de créer la possibilité de faire fonctionner ces trop grandes intercommunalités. Mais, dans certains cas, ça ne suffit pas ! Alors, que faut-il faire ? Maintenir à toute force unies par les liens de l'intercommunalité des communes qui ne réussissent pas à travailler ensemble, ou tirer les conséquences de leur mésentente en essayant de construire quelque chose d'autre, qui relève toujours, d'ailleurs, de l'intercommunalité ? Car on a tort de vouloir opposer communes et intercommunalité ! L'intercommunalité est un instrument nécessaire pour toutes les communes. Recherchons, là où vraiment toutes les alternatives auront été épuisées, la possibilité de modifier à la marge, dans des cas exceptionnels, la carte intercommunale, et créons des procédures en

Cette possibilité n'existe que par décision du préfet ! Or nous préférons la décision de la commission départementale de la coopération intercommunale à celle du préfet ! Pourquoi ? Parce que c'est plus démocratique ! Et nous préférons, nous, toujours, faire confiance aux élus plutôt que de demander au préfet de se faire le juge du divorce. Les parties doivent réussir à trouver une solution